Madame la ministre, mes chers collègues, par lettre en date du 21 novembre 2017, le Gouvernement a demandé l'inscription à l'ordre du jour du mardi 19 décembre des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, ou de sa nouvelle lecture, après l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2018, ou de sa nouvelle lecture. Acte est donné de cette demande. Nous pourrions prévoir une discussion générale commune d'une heure pour ces deux textes. Y a-t-il des observations ? observations ? ... Il en est ainsi décidé. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018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

Mes chers collègues, je vous rappelle que les deux premiers débats que nous allons tenir cet après-midi sont inscrits dans l'espace réservé d'un groupe politique.

à respecter scrupuleusement son temps de parole. La formule choisie pour ces débats est intéressante, mais elle nécessite beaucoup de discipline

rapporteur pour la commission des lois, pour son travail, même si Alain Bertrand eût préféré examiner une proposition de loi, ce qui était son projet initial. J'aimerais vous présenter les motifs de la présentation de cette proposition de loi, que nous avons accepté de transformer en débat. Plusieurs maires et maires délégués nous ont saisis, dans nos territoires, du problème de la représentativité à long terme des communes déléguées au sein des communes nouvelles. Pour les élections municipales prévues en 2020, il est prévu une baisse importante du nombre de conseillers municipaux des communes nouvelles, ce qui suscite une certaine inquiétude chez les élus locaux. Dans les chartes de communes nouvelles, cette représentativité des communes déléguées est souvent exprimée. Pour autant, elle ne revêt aucun caractère obligatoire, ce qui relativise cette représentativité. Les effets sur l'effectif du conseil municipal de la commune nouvelle sont lissés dans le temps. Dans un premier temps, entre la création de la commune nouvelle et le renouvellement du conseil municipal, c'est-à-dire, pour les communes nouvelles déjà créées, jusqu'en 2020, territoriales dispose : « Jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé [ ...] de l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes de la deuxième période transitoire, entre 2020 et 2026, pour les communes nouvelles déjà créées, s'appliquera l'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, dispose : « [ ...] Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l'article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. » Enfin, à partir de 2026, pour les communes nouvelles déjà créées, le nombre de conseillers sera encore réduit

Lors des prochaines élections municipales de 2020, rien n'obligera donc les listes candidates à comporter des représentants de chacune des communes déléguées formant la commune nouvelle. De même, en cas de démission ou de décès du maire délégué, seul représentant de sa commune initiale, la représentativité ne sera pas assurée, à partir de 2020, si aucune personne sur la liste n'appartient à la même commune déléguée. Ce manque de pérennité de la représentativité territoriale a un effet bloquant pour les petites communes qui envisagent d'intégrer ou de créer une commune nouvelle. une loi qui assurerait la pérennité de la représentation des communes déléguées permettrait l'aboutissement de nombreux projets de communes nouvelles, les ruraux souhaitant se regrouper et refusant, en revanche, de voir disparaître l'histoire et le patrimoine culturel de leurs anciennes communes, auxquels il est bien normal notre groupe, en particulier Alain Bertrand, ont donc pris l'initiative de rédiger la proposition de loi visant à garantir la représentation des communes déléguées au sein des communes nouvelles. dans sa rédaction initiale, pour les communes de plus de 1 000 habitants, trois conséquences majeures. Premièrement, la liste des candidats à la commune nouvelle devrait être composée de candidats résidant dans chaque commune déléguée. Deuxièmement, le maire délégué devrait être choisi parmi les conseillers municipaux résidant dans la commune déléguée. Troisièmement, un conseiller municipal décédé ou démissionnaire ne pourrait être remplacé que par un candidat résidant dans la même commune déléguée que lui. De plus, des maires et maires délégués, ainsi que plusieurs collègues sénatrices et sénateurs, nous ont fait remarquer qu'il serait injuste d'appliquer ce dispositif aux seules communes nouvelles de plus de 1 000 habitants. Le problème est que les conseillers municipaux dans les villes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin majoritaire, conformément à l'article L. 252 du code électoral. Avec ce type de scrutin, il est impossible de garantir sur le long terme la représentativité des communes déléguées, puisque l'ordre de la liste peut être modifié par les électeurs. La seule solution, à mes yeux, serait d'appliquer le scrutin de liste à toutes les communes nouvelles, peu importe leur nombre d'habitants. C'était l'objet

commission par la commission des lois. Je voudrais à présent revenir sur plusieurs observations faites par Mme la rapporteur à Alain Bertrand, lors de son audition, avant la rédaction de son rapport. Mme la rapporteur insiste sur le fait que la création de communes nouvelles a d'abord pour origine une démarche volontaire des élus, désireux de bâtir ensemble un nouveau destin. Si nous pouvons être en accord avec ces propos, nous tenons tout de même à préciser qu'avoir un projet commun, vouloir construire ensemble, n'empêche nullement les communes déléguées de souhaiter garder leur identité et s'assurer de la représentation de leur histoire et de leur ancien statut

Note collègue a notamment précisé que, selon elle, comme il était dans l'intérêt des candidats aux municipales de constituer des listes avec des représentants de tous les quartiers, donc de toutes les communes déléguées, la représentation serait assurée naturellement,

qu'il pourrait en être autrement dans les faits. Imaginons quatre petites communes A, B, C et D qui souhaitent constituer une commune nouvelle. La commune A compte 900 habitants et les communes B, C et D ont 50 habitants chacune, ce qui ferait un total de 1 050 habitants pour la nouvelle commune.

il n'y a aucun intérêt, ou impératif stratégique électoral, pour les candidats issus majoritairement de l'ancienne commune A, la plus importante, de laisser des places éligibles sur leur liste à des candidats issus des communes B, C et D.

Le bon sens rural les pousse, car ils connaissent bien les faiblesses de la nature humaine, à demander des garanties sur la représentation historique, patrimoniale et culturelle, fonctionnelle même, afin de garantir leur avenir au sein de la commune nouvelle. Leur demande est ordinaire et légitime. Je ne prétends pas que notre texte était parfait, mais nous aurions pu probablement ensemble, avec un peu de bonne volonté, trouver les moyens de l'améliorer. Pour autant, nous pouvons nous satisfaire qu'il soit l'occasion de lancer le débat, et que chacun d'entre nous reconnaisse qu'un ajustement du régime juridique des communes nouvelles est nécessaire, et cela rapidement, avant 2020. La création d'une commune nouvelle ne signifie pas la disparition des prérogatives et des droits attachés au passé et à la formation de l'avenir, pour certaines parties de territoire. Ce serait contraire à l'esprit même qui préside à la création des communes nouvelles

qu'en l'état actuel de la loi certaines communes déléguées ne pourraient pas être représentées dans la commune nouvelle : « Dans certains cas il n'y aurait pas assez de sièges à pourvoir pour assurer la représentation de l'ensemble des communes déléguées.

de liste résidant dans la même commune, ou l'élection du maire délégué parmi les élus de la commune déléguée, tombent sous le sens et peuvent être prévus par quelques ajustements juridiques. Au total,

ce débat est l'occasion de revenir sur un sujet qui est cher au Gouvernement : les communes nouvelles. Les échanges que nous menons sur l'ensemble des sujets relatifs aux collectivités territoriales dans le cadre de la Conférence nationale des territoires ne peuvent qu'être nourris par des initiatives comme les communes nouvelles, qui donnent vie au débat et corps aux ambitieux projets locaux portés par les élus. Les communes nouvelles sont l'un des symboles de ce qui marche dans nos territoires, et sont le gage d'une meilleure administration et de meilleurs services rendus à la population, là où les élus le souhaitent. Permettez-moi d'ajouter que l'État a été, sur cette question des communes nouvelles, un partenaire attentif, soucieux de faciliter et d'accompagner des initiatives dont il perçoit les avantages évidents pour l'action publique sur les territoires qui se l'approprient.

pour des communes fortes et vivantes, qui a permis d'asseoir le succès de cette réorganisation territoriale. Ce dernier texte avait d'ailleurs été inspiré par l'AMF, l'Association des maires de France,

par son caractère d'exercice parfois imposé, susciter des réactions de la part des élus, les communes nouvelles reposent entièrement sur l'initiative et la libre volonté des communes. communes. Ce système a permis à 1 760 communes de fusionner pour former 517 communes nouvelles- 317 jusqu'au 1 janvier 2016, et 200 entre le 2 janvier 2016 et le 1 janvier 2017 rassemblant une population totale de près de 1,8 million d'habitants, ce qui faisait ainsi passer la France sous le seuil symbolique des 36 000 communes avec 35 498 communes au 1 janvier 2017.

Le Gouvernement croit cependant toujours en la force du modèle proposé par les communes nouvelles et compte accompagner son développement.

aux communes de moins de 1 000 habitants et à celles de 10 000 à 15 000 habitants. Jusqu'à présent, la mesure s'appliquait seulement aux communes nouvelles de 1 000 à 10 000 habitants ; un amendement adopté à l'Assemblée nationale a supprimé le seuil et a rehaussé le plafond de 10 000 à 15 000 le soutien à l'investissement local sera stabilisé pour l'ensemble des collectivités territoriales et un fonds de modernisation de 50 millions d'euros sera créé au sein de la dotation de soutien

communes nouvelles. La procédure améliorée pour la graphie des noms des communes nouvelles, une circulaire du 18 avril 2017.

est prévue la dérogation à l'application de la parité pour l'élection des adjoints, dans certaines conditions et de façon transitoire, dans les communes de plus de 1 000 habitants issues de la fusion de communes anciennes de moins de 1 000 habitants.

d'une part, à l'esprit qui vise à faire de la commune nouvelle une véritable commune et, d'autre part, aux principes constitutionnels. Le critère de résidence dans la commune déléguée porte différenciation entre les candidats et constitue ainsi une rupture d'égalité devant le suffrage.

Pour rappel, lors de sa création et jusqu'au prochain renouvellement, le conseil municipal de la commune nouvelle peut être composé de la somme des conseillers des anciennes communes, puis il bénéficie de la strate démographique

Cette proposition pérennise le dispositif dérogatoire, tandis que le Gouvernement soutient que les communes nouvelles sont des communes à part entière. Je ne peux pas le dire plus simplement. Je

sans une volonté commune autour d'un projet d'avenir, et d'une vision partagée du territoire coconstruit avec les acteurs locaux et soutenue par tous ». Ce sont également les conclusions des premières Assises nationales des communes nouvelles, organisées par l'AMF, auxquelles j'ai eu le plaisir de participer le 12 octobre dernier.

Vous l'avez rappelé, madame la ministre, entre 2015 et 2016, et du fait de l'unique volonté des élus locaux, le tissu communal a connu une rationalisation sans précédent : plus de plus de 500 communes nouvelles ont été créées, représentant 1 800 communes historiques et 25 000 conseillers municipaux, 1,7 million de nos concitoyens étant concernés. nos concitoyens étant concernés. Vous noterez que cette transformation inédite du paysage communal est la preuve de la capacité d'adaptation et d'innovation des territoires, dès lors que la souplesse du régime juridique permet de respecter les spécificités territoriales. En matière de gouvernance, 95 % des communes nouvelles ont opté pour le régime dérogatoire et transitoire permettant d'augmenter le nombre de conseillers municipaux. Par ailleurs, 95 % de ces communes ont choisi de créer des communes déléguées. Le prochain renouvellement général, celui de 2020, suscite des inquiétudes légitimes chez les élus locaux quant à la représentativité des communes fondatrices. Il marquera en effet la fin de ce régime dérogatoire, ce qui se traduira par une diminution brutale, de 50 % en moyenne mais

Vous l'avez dit, les communes nouvelles constituent bien de nouvelles entités, de nouvelles communes, et non une supracommunalité. Néanmoins, l'objectif est de faire en sorte d'assurer la meilleure représentativité possible de toutes ces composantes sans pour autant ajouter de la complexité à un système qui repose avant tout sur la souplesse et la volonté des élus. Dans cette optique, la possibilité du caractère obligatoire de la charte de la commune nouvelle, aujourd'hui facultative, peut-elle être examinée ? revisité avant chaque fin de mandat, demeurerait régi par des principes de souplesse pour que chaque commune nouvelle définisse sa propre gouvernance et garantisse la représentativité des communes historiques. La parole

les supports de la réflexion et des conclusions de travail ayant amené à la création de la commune nouvelle. Cette charte

touchant à la réglementation et qui ne seraient pas acceptables juridiquement, car la loi précise déjà beaucoup de choses sur la création et l'organisation des communes nouvelles. Ensuite, je crois que cela alourdirait le fonctionnement des communes nouvelles.

au 1 janvier 2017, issues de la fusion de 1 760 communes, comptent aujourd'hui 24 139 conseillers municipaux. Cette démarche volontaire des élus a été encouragée non seulement par un pacte financier, mais aussi par la faculté de conserver les communes historiques sous forme de communes déléguées. Pour faciliter la création de communes nouvelles, un régime dérogatoire au droit commun permet d'augmenter à titre transitoire l'effectif de leurs conseils municipaux et donne ainsi la possibilité aux élus des communes historiques d'y siéger.

et d'environ 56 % en 2026, selon les estimations de l'AMF. Cette baisse, parfois brutale, engendre, chez les élus qui ont mis en place des communes nouvelles comme chez ceux qui envisagent de le faire, la crainte d'une représentation insuffisante de certaines communes déléguées au conseil municipal de la commune nouvelle.

l'addition des représentants à la strate supérieure puis à la strate de la population. Je ne peux rien vous dire de plus que

tout de même quelques points. Les anciennes communes deviennent toutes automatiquement des communes déléguées, sauf décision contraire des conseils municipaux prise avant la création de la commune nouvelle. nouvelle. Le plafonnement du nombre d'adjoints au maire à 30 % de l'effectif légal du conseil municipal est aménagé, puisque la loi du 16 mars 2015 prévoit que les maires délégués exercent également les fonctions d'adjoint au maire

délégué et d'une annexe de la mairie, dans laquelle sont établis les actes d'état civil concernant les habitants de la commune déléguée. Le maire délégué est officier d'état civil et de police judiciaire de la commune déléguée ; il peut, par ailleurs, recevoir des délégations territorialisées de la part du maire de la commune nouvelle. Il est également possible de créer un conseil de la commune déléguée, composé d'un maire délégué et de conseillers municipaux, sur décision du conseil municipal de la commune nouvelle statuant à la majorité des deux tiers de ses membres. Le conseil municipal d'une commune nouvelle peut également instituer une conférence municipale présidée par le maire et comprenant des maires délégués, au sein de laquelle peut être débattue toute question de coordination de l'action publique sur le territoire de la commune nouvelle. Le rapport entre la commune nouvelle et ses communes déléguées est donc vraiment souple, libéral, et il respecte les particularités des communes historiques.

associées, je souhaite soulever deux écueils qui doivent être évités dans la représentation des communes déléguées au sein des communes nouvelles. Le premier écueil à donner l'illusion du maintien d'une démocratie de proximité en maintenant une représentation à long terme des communes déléguées au sein des communes nouvelles, à l'image des communes associées de la loi du

Reprenant la célèbre formule de ma collègue Françoise Gatel, je dirais que, pour moi, une commune nouvelle est une nouvelle commune ; elle doit permettre à terme l'intégration totale de l'ensemble de ses composantes.

rapprochement des communes, et sur la volonté de travailler ensemble. Chaque commune nouvelle a ses spécificités qui doivent être maintenues. On doit faire confiance aux élus locaux pour mettre en place les conditions de l'intégration et de la représentation de l'ensemble des territoires, qui sont garants

et ne pas entrer dans un système de normes réglementaires, qui rigidifieraient le système et qui empêcheraient la création de communes nouvelles

avant d'entrer dans le vif de mon interpellation, il me paraît important de préciser un point fondamental. Nous ne devons pas oublier que les communes déléguées n'ont pas vocation à s'ancrer dans le temps. Bien au contraire, elles ne sont qu'un instrument permettant une progression plus tranquille entre le groupement de communes et la commune nouvelle formée. C'est cette perspective qui doit conditionner nos raisonnements. tout dispositif visant à renforcer leur représentation au sein des communes nouvelles doit être mûrement réfléchi ; il ne doit pas entraîner de rigidité trop importante, il ne doit pas faire de la commune déléguée une sous-commune ayant des fonctions autres que celle qui consiste à assurer une période de transition progressive et fluide et à garantir un lien de proximité un lien de proximité avec les habitants. Inciter à la création de communes nouvelles garantit justement une certaine souplesse. À cet égard, nous pourrions justement réfléchir aux moyens d'ancrer dans le dispositif législatif le caractère intrinsèquement péremptoire de la commune déléguée, afin qu'il soit établi plus clairement que, si elles garantissent un lien de proximité étroit avec les habitants, elles n'ont pas vocation à durer dans le temps. La législation en vigueur dispose que le « conseil municipal peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu'il détermine. On ne saurait imaginer une commune nouvelle prospérant avec, en son sein, des communes déléguées existant pour une durée parfaitement indéterminée. Madame la ministre, quelle est votre position sur le sujet, et quel dispositif peut être, selon vous, afin de concilier la souplesse et la clarté que sollicite la législation sur ce point ? D'abord, je suis globalement d'accord avec ce que vous venez de dire. Ce sont des

fin du débat. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Il est des communes nouvelles de bon sens ; il en est au moins autant qui sont nées d'un réflexe de défense contre la pénurie financière,

Il en est aussi qui ont été abusées par l'illusion entretenue que les mesures temporaires permettant la survie symbolique des communes dans la commune nouvelle seraient éternelles. Beaucoup découvrent aujourd'hui qu'il n'en est rien ; toutes les dispositions incitatives n'y changeront rien. Ma question est la suivante : pourquoi ne pas répondre à leurs attentes ? Qu'est-ce qui s'y oppose ?

si je puis dire, dans les habitudes de travailler ensemble. Je ne peux pas aller plus loin dans le raisonnement ; autrement, on n'atteindrait pas le but que l'on s'est fixé au départ, que se sont fixé

Madame la ministre, je constate que ce qui est permis aux métropoles devient une anomalie inacceptable pour ce qui concerne les petites communes. Une commune nouvelle n'est pas un EPCI, dites-vous, mais un EPCI, en revanche, peut cacher une commune qui ne dit pas son nom. Je pense, par exemple, à la métropole lyonnaise. Ils étaient partis pour faire un EPCI, ils se retrouvent avec une commune

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, mon propos va plutôt porter sur les bonnes conditions de mise en oeuvre du territoire vécu ; c'est un élément aussi prégnant pour l'avenir de la commune nouvelle que celui de la représentation. Avec la refonte territoriale, 517 communes nouvelles ont vu le jour- c'est un succès, on peut le dire -, et on en compte 37 dans le Calvados. Cette refonte bouscule nos habitudes, nos frontières du quotidien et il ne faut pas oublier que le succès des communes nouvelles a été garanti par les élus locaux qui ont veillé chaque fois à une organisation adaptée aux spécificités de leur territoire et de leurs habitants. Cela s'est fait aussi, bien sûr, sur le fondement d'engagements financiers et contractuels de l'État, qui ont accompagné ce mouvement des communes nouvelles et qui conditionnent leur avenir. Pour faciliter l'ancrage de la commune nouvelle, l'État doit veiller- cela a d'ailleurs souvent été le cas -à reconduire les agréments et les aides obtenus préalablement par les communes historiques.

Or ces sujets ont conditionné en grande partie la nature des engagements consentis entre communes historiques pour réaliser le projet de territoire de leur commune nouvelle. Le coeur de tout cela est bien que, en vivant au quotidien la commune nouvelle, les habitants s'emparent de leur nouveau territoire et, pour cela, il faut un peu de stabilité.

Dans ces conditions, ne pourriez-vous envisager un délai de trois ans, comme le préconisait judicieusement le rapport de nos collègues Françoise Gatel et Christian Manable ? Ces trois ans donneraient le temps au projet de s'exprimer avant de modifier les agréments et les engagements de l'État qui avaient permis au projet d'origine de la commune nouvelle de réaliser un territoire cohérent.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le département de Maine-et-Loire est fortement marqué par le phénomène de regroupement de communes, puisqu'il compte actuellement 34 communes nouvelles. Au 1 janvier 2017, il y avait 186 communes contre 358 en 2015, soit près de la moitié de communes en moins ! Les élus d'Anjou ont manifestement réussi à dépasser les clivages partisans et à faire passer l'intérêt collectif avant l'esprit de clocher. Vous les avez d'ailleurs rencontrés dans un esprit d'ouverture, lors d'une table ronde au mois de juillet dernier. Je souhaite ici saluer le soutien apporté à cette dynamique dans le projet de loi de finances pour Même si le seuil de 10 000 habitants est discutable, le maintien de la DGF et la bonification de 5 % de la dotation forfaitaire pour les communes nouvelles sont une bonne chose. très instructif de nos collègues, ici présents, Christian Manable et Françoise Gatel, sur la « révolution silencieuse » des territoires avait repéré, dès 2016, un ensemble de points qui restaient à améliorer et qui demeurent d'actualité. En augmentant la taille de sa population, la commune nouvelle peut être soumise à de nouvelles obligations en matière de construction de logements sociaux ou d'accueil des gens du voyage.

Ce besoin de temps est également évoqué par les élus pour l'établissement de documents d'urbanisme communs ou encore pour la création d'un centre communal d'action sociale, la construction d'écoles ou la création de comités techniques paritaires. Cette période de transition peut paraître trop courte pour des territoires ruraux, qui demandent une prise en compte des spécificités du terrain. J'en arrive à ma question : le Gouvernement envisage-t-il des mesures d'accompagnement renforcé pour ces communes nouvelles, afin qu'elles puissent s'adapter à temps à leurs nouvelles obligations ? La parole est à Mme la ministre. Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur les nouvelles obligations s'imposant aux communes nouvelles franchissant un seuil de population en matière de construction d'aires d'accueil des gens du voyage- plus de 5 000 habitants

La pénalisation financière concernant les logements sociaux ne s'applique pas les trois premières années et permet donc aux communes nouvelles d'engager des projets. Nous le savons, la demande de logements, plus particulièrement de logements sociaux, est forte dans le pays.

En Marche. Madame la ministre, la fin de la période de transition prévue par le régime juridique des communes nouvelles suscite de nombreuses inquiétudes auprès des élus locaux, en raison de la diminution progressive de l'effectif des conseils municipaux des communes communes nouvelles. En l'état du droit, la représentation des communes déléguées au sein des communes nouvelles à l'occasion des prochains renouvellements n'est, en effet, ni organisée ni obligatoire. Pour autant, l'introduction de contraintes spécifiques dans la constitution des listes municipales en fonction du lieu de résidence des candidats conduirait à une rigidité excessive et méconnaîtrait la philosophie sous-jacente à la création des communes nouvelles. Au contraire, il faut continuer d'encourager les élus impliqués à bâtir des communes nouvelles à partir de projets de territoire ambitieux. Dans cette optique, madame la ministre, serait-il envisageable de modifier l'article 7 de la loi 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux, qui implique, afin d'éviter les redécoupages électoraux tardifs, qu'aucune commune nouvelle ne pourra être créée à compter de mars 2019 ? Mon collègue Arnaud de Belenet a ainsi par amendement, de prendre en compte la date de prise de l'arrêté créant la commune nouvelle plutôt que sa date d'effet, afin de pouvoir créer une commune nouvelle au 1 janvier 2020, dès lors que l'arrêté serait pris avant mars 2019. Nous souhaiterions connaître l'avis du Gouvernement sur cette proposition, qui est assurément de nature à encourager la création de communes nouvelles, en allant dans le sens de l'action gouvernementale. est à Mme la ministre. Madame la sénatrice, chère Patricia Schillinger, vous proposez de permettre la création de communes nouvelles jusqu'au 1 janvier 2020, soit quelques semaines avant le renouvellement général des conseils municipaux et donc de déroger aux dispositions de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990, qui prévoit qu'« il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées. Si, dès 1990, le législateur a prévu une année blanche dans le redécoupage des circonscriptions électorales avant l'échéance normale de renouvellement, c'est avant tout dans un souci de lisibilité pour les électeurs. En effet, le délai d'un an garantit à nos concitoyens de connaître précisément le ressort territorial de l'élection à venir. Permettre la création de communes déléguées jusqu'au 1 janvier 2020 aurait pour conséquence que les électeurs concernés votent dans un ressort créé seulement trois mois auparavant. Je veux par ailleurs rappeler que le projet de loi de finances pour 2018 prévoit une réactivation du dispositif de maintien de la DGF pour les communes nouvelles créées au plus tard au 1 janvier 2019, en s'appuyant, bien sûr, sur les calendriers actuels. Dans ces conditions et pour toutes ces raisons, il ne nous paraît pas opportun de revenir sur l'existence de cette année blanche, garantie de lisibilité pour nos concitoyens, mais aussi pour ceux qui envisagent de se présenter aux élections sur un territoire municipal. La parole est

et près de 1,8 million d'habitants. La mise en place d'un assouplissement du régime juridique a participé à l'essor de ces rassemblements de communes, tout comme la création du statut de commune déléguée, qui a permis aux communes ayant fusionné à la fois de conserver leur propre identité historique et de mettre en commun leurs moyens. Cependant, nous sommes en droit de nous interroger sur la finalité de ces communes déléguées, comme l'ont fait d'autres interlocuteurs avant moi. Il paraît tout de même illusoire de donner à penser aux maires des futures communes déléguées que leur commune survivra à la fusion après 2020. Il faut, bien au contraire, faire preuve de transparence et d'honnêteté intellectuelle. Ne nous y trompons pas : la fusion vise, à terme, à réunir des communes au sein d'une nouvelle commune, qui englobera définitivement les anciennes communes après une période de transition définie, en outre le rôle des communes déléguées. Dès lors, la question de la représentation de ces communes déléguées au sein des communes nouvelles doit être clarifiée. Il doit s'agir d'une démarche volontaire des élus locaux. Ceux-ci doivent recevoir toutes les informations sur l'avenir de leur commune devenue déléguée et vouée, de fait, à disparaître à terme. Les incitations financières de l'État ne semblent pas aller dans ce sens. Pourquoi maintenir les incitations fiscales s'il s'agit d'un choix local et d'une démarche libre ? L'argumentation idéologique sous-jacente repose, bien entendu, sur la diminution du nombre de communes et sur un alignement de notre pays sur les autres modèles européens. Aussi, madame la ministre, que comptez-vous mettre en place pour que chaque maire ayant à prendre la décision d'intégrer ou non sa commune au sein d'une commune nouvelle ait tous les éléments objectifs à sa disposition afin de pouvoir faire un choix éclairé sur le devenir de sa commune, sans avoir à se fonder uniquement sur les avantages financiers proposés ?

je sais que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais je crois que l'esprit

peu moins ... Mon collègue Christian Manable et moi-même avons eu l'occasion de constater la révolution silencieuse qu'est la création de communes nouvelles, qu'il convient de faciliter. J'ai moi aussi une proposition très précise à formuler, non pas pour remettre en cause le principe général, mais pour faciliter la création des communes nouvelles : elle consiste à allonger la période transitoire,

à trois fois le nombre de leurs communes, soit, pour La Hague, 57 conseillers municipaux au lieu de 35, ce qui est un élément facilitant pour la création de communes nouvelles, qui va devenir un exercice difficile, un an avant les élections. La parole est à Mme la ministre.

La parole est à M. Christian Manable, pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'essor récent des communes nouvelles marque un tournant riche d'enseignements.

Le succès de ces regroupements est dû à la conception même de la loi du 16 mars 2015, largement inspirée par les débats au sein de l'Association des maires de France. Je veux insister sur les termes conçu par et pour le terrain » : le mouvement a été amorcé par les élus eux-mêmes, sur la seule base du volontariat. Or, si le succès des communes nouvelles est réel, il n'est pas uniforme en France. Alors que certains départements comptent jusqu'à 36 communes nouvelles créées au 1 janvier 2017, comme c'est le cas de la Manche, le meilleur exemple reste toutefois le Maine-et-Loire, dont près de 50 % de 360 communes se sont regroupées,

C'est parfois dans les départements qui en auraient le plus besoin, où se trouvent plusieurs communes rurales isolées, dépeuplées et sans moyens, que les chiffres sont décevants.

D'ailleurs, dans les départements où le nombre de communes nouvelles est important, on constate une action importante de la part des services de l'État. Madame la ministre, j'en viens à ma question,

assez largement recours à ce nouvel instrument qu'est la commune nouvelle, que l'Association des maires de France avait voulu mettre en place. Aujourd'hui,

et avec des compétences d'autant plus grandes que certaines de ces grandes intercommunalités rurales ont le statut de communauté d'agglomération, comme s'il s'agissait de grands territoires urbains. Si nous voulons, demain, à la fois faire réussir ces très grandes intercommunalités et préserver la vitalité de la commune comme cellule de base de la démocratie, il faut trouver le bon équilibre entre l'infiniment grand et l'infiniment petit.

des communes nouvelles se sont naturellement créées pour entrer ou pour peser davantage dans les grandes intercommunalités. Cela a été l'une des raisons

La parole est à M. Jean-Marie Janssens, pour le groupe Union Centriste. Madame la ministre, depuis la réforme territoriale de 2010 et la création du statut de commune nouvelle, plus de 500- 517 exactement -communes nouvelles ont été créées en France, regroupant près de 2 millions d'habitants. On le voit, le modèle communal français est en mutation. Oui, la France des 36 000 communes a vécu. Cette réalité ne signifie pas la mort des petites communes et de l'action de proximité. Au contraire, la commune est et doit rester le socle et le ciment de notre République française. Pour cela, il faut que les communes nouvelles soient valorisées dans leur rôle de protectrices de l'action locale de proximité. d'encourager les communes à se regrouper en communes nouvelles, l'État a mis en place un dispositif d'incitation financière en 2015. Un pacte financier n'est cependant pas suffisant. Ce que nous réclamons, nous, les représentants des communes, c'est un vrai pacte de proximité passé entre l'État et les communes nouvelles, oui, un pacte qui garantisse aux communes nouvelles le maintien des services publics de proximité et des services de l'État, la sanctuarisation des dotations de l'État, à commencer par la DETR, indispensable à l'investissement local, l'aide au maintien des commerces, un accompagnement dans la revitalisation des bourgs, un soutien efficace dans la lutte contre la baisse de la démographie médicale. Tout cela est particulièrement nécessaire dans les territoires ruraux, qui traversent de grandes difficultés financières et démographiques. Ce pacte de proximité doit être plus qu'une incitation. Il doit consacrer la relation de confiance qui unit l'État aux communes, quelle que soit leur taille. Madame la ministre, pouvez-vous nous assurer aujourd'hui que l'État ne se désengagera pas vis-à-vis des communes et qu'il continuera à encourager la création de communes nouvelles en leur offrant des garanties durables en matière de services publics de proximité ? La parole est à Mme la ministre.

la clause de compétence générale est maintenue au seul niveau de la commune et que, naturellement, l'État doit accompagner les communes nouvelles comme toutes les communes de France, pour que les services publics soient assurés. Si j'ai bien compris votre raisonnement,

pour le groupe socialiste et républicain. La « commune nouvelle » apparaît dans notre paysage institutionnel comme une nouvelle forme d'organisation susceptible, pour les élus qui ont voulu s'en saisir, de répondre de façon plus efficiente aux besoins de leur population. Ce débat nous amène à repenser la place de la commune dans la République. Je suis de ceux pour qui la commune doit rester l'entité de base de notre démocratie républicaine, et ce pour trois raisons au moins.

Elle doit même les rendre possibles, les conforter. Alors que la plupart des élus locaux vivent très mal- et ils nous le disent ! -le déclassement de la commune et l'expression au plus haut niveau d'un dédain à l'égard de leur engagement bénévole-

Le jour où ce sera le cas, il en sera terminé des communes ! Exactement ! Les « communes nouvelles » ont-elles vocation à se substituer aux communes à la faveur, par exemple, de mécanismes financiers qui obligeraient, sans le dire, et c'est déjà le cas, les communes à se regrouper ?

La France est une République une et indivisible. On agit toujours dans le cadre de la loi, on ne peut pas faire n'importe quoi.

la loi dite Marcellin a permis, dans certains départements, la création de nombreuses communes dites « associées », théoriquement sur la base du volontariat. En réalité, elles le furent sous la pression, certes bienveillante, mais très présente, des préfets. En Haute-Marne, par exemple, plus de 200 communes

? C'est là tout le fond de ma question. Désormais, avec l'accord du conseil municipal, les anciennes communes associées peuvent se voir reconnaître le statut de commune déléguée. Alors que le Gouvernement appelle à une réduction globale du nombre d'élus, pourtant quasiment bénévoles en milieu rural, pouvez-vous garantir, madame la ministre, que vous n'avez pas l'intention de faire disparaître les communes déléguées dans la discrétion et l'indifférence quasi générale, comme vos prédécesseurs ont essayé de le faire avec les communes associées ? La parole est à Mme la ministre. Non, monsieur

permet parfois de rester dans une structure unique. Il n'y a toutefois aucune volonté particulière de faire disparaître les communes déléguées. Je me souviens très bien de la manière dont vous avez déposé ce texte pour faciliter l'entrée des communes « Marcellin » dans le système des communes nouvelles, ce qui était bien sûr une très bonne idée. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le débat que nous avons aujourd'hui est très instructif, alors que se déroule, à quelques pas de notre hémicycle, le centième congrès des maires de France. Je tiens d'ailleurs à remercier nos collègues qui nous offrent cette opportunité. La dynamique du regroupement des communes est une réalité. On compte, dans bon nombre de nos départements, des initiatives qui ont- ou vont -aboutir à des communes plus peuplées et, par conséquent, plus fortes. En effet, avec des communautés de communes de taille parfois « XXL », la commune nouvelle peut constituer une réponse adéquate pour peser davantage dans les prises de décisions communautaires. Pour en parler régulièrement avec les maires qui ont franchi le pas, et dont je salue le courage et l'audace, nous savons tous que les communes nouvelles ne sont synonymes de réussite que si elles s'inscrivent dans un projet de territoire. Et qui dit projet entend plus de services publics, plus d'équipements et, donc, plus d'investissement ! Si, à l'avenir, les communes nouvelles sont celles qui sont les plus dynamiques, je ne pense pas que la question de la représentation des communes déléguées au sein des communes nouvelles constitue un sujet de préoccupation principal pour les élus locaux ou un frein à la mise en oeuvre de ces dernières. La loi du 16 mars 2015 prévoyait des garanties de ressources pour les communes nouvelles créées avant le 1 janvier 2016. Un dispositif permettait à ces communes de bénéficier du gel de la DGF et de certaines bonifications, ou de gels de dotation, comme la DSR. Ce dispositif a été prorogé jusqu'au 1 janvier 2017. Si l'on veut encourager de nouveaux rapprochements, l'État doit accompagner les projets de création ou d'extension de communes. Un nouveau pacte de stabilité de la DGF et une dotation spécifique aux communes nouvelles pourraient être une réponse adaptée, notamment dans les territoires ruraux et de montagne, où le potentiel est important. C'est pourquoi, madame la ministre, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer si de nouvelles mesures seront envisagées à partir du 1 janvier 2018. La parole est à Mme la ministre. Oui, madame la sénatrice Morhet-Richaud,

Bien évidemment, la DGF étant répartie au sein d'une enveloppe normée, vous comprenez que nous fixions un plafond.

madame la ministre, participé à leurs travaux. À cette occasion un premier bilan a pu être fait de l'application de la loi du 16 novembre 2015, confirmant le succès des assouplissements et des incitations apportés à ce dispositif. Celles et ceux qui m'ont précédé ont rappelé les chiffres : ils témoignent d'une tendance que nous ressentons également sur le terrain. Toutefois, nous devons sans cesse rappeler qu'une commune nouvelle doit être appréhendée comme une nouvelle commune. nous devons dire aux élus souhaitant s'engager dans la création d'une commune nouvelle qu'elle est une fusion, pas une intercommunalité, ni une coopération de proximité. Cela permettra de se prémunir de certaines déconvenues que nous voyons poindre. En outre, au sein de ces nouveaux ensembles, le respect des identités des communes déléguées est primordial. C'est une question de représentativité démocratique. L'avenir du fait communal dépend aujourd'hui de sa capacité à se rénover. L'évolution des communes nouvelles est une des manifestations du dynamisme de cet échelon.

Je pense notamment à celles exposées en matière d'évolution de l'effectif du conseil municipal et concernant la création d'une dotation temporaire spécifique commune nouvelle. La parole est à Mme

L'ordre du jour appelle le débat,

et républicain, disposera d'un temps de parole de dix minutes, y compris la réplique, puis le Gouvernement répondra pour une durée qui ne

nul ne doute aujourd'hui de l'extrême importance des enjeux énergétiques pour l'avenir de nos sociétés. Il s'agit tout d'abord de répondre aux enjeux de la crise climatique, très liée aux consommations fossiles. Ce défi est redoutable, tant il y va de l'avenir même, au XXI siècle, de nos sociétés, dont nous savons qu'elles ne survivront pas aux crises alimentaires et migratoires mondiales qu'engendrerait un réchauffement supérieur au seuil d'augmentation de 2 degrés que la communauté scientifique nous fixe comme limite d'acceptation pour la résilience de nos sociétés. Il faut aussi, dans le monde économique classique qui continue de rythmer notre quotidien, tenir compte des enjeux de sécurité d'approvisionnement et de distribution, respecter la solidarité entre territoires, lutter contre les précarités et maintenir une économie compétitive dans un monde économique libéral- cette liste n'est probablement pas exhaustive. Construire une stratégie énergétique nationale cohérente, intégrant tous ces enjeux, mariant court et long termes, tenant compte des capacités d'investissements publics et privés et s'inscrivant dans le cadre européen n'est pas chose totalement aisée, nous n'en disconvenons pas. le groupe du RDSE aime les défis intellectuels, ... Très bien ! ... et nous ne doutons pas que ces deux heures de discussion contribueront utilement à alimenter la réflexion et à nourrir le travail de préparation de la programmation pluriannuelle de l'énergie

Je n'ai donc pas, dans le cadre de cette introduction, la prétention de proposer un plan exhaustif de la transition à mener- nous avons encore quelques mois de discussion devant nous -, mais je voudrais insister sur quelques points. Le groupe du RDSE, à l'origine de ce débat par l'intermédiaire de notre collègue Raymond Vall, que je salue, a une réputation de diversité, qu'il assume. Et il est vrai que, s'agissant par exemple du regard porté sur l'énergie nucléaire, quelques légères nuances peuvent exister entre nous. Mais les échanges que nous avons eus, depuis deux mois, au sein de notre groupe ont surtout témoigné de l'existence de nombreuses réflexions communes, à partir d'une acceptation collective de la nécessité de s'engager résolument dans une transition énergétique devenue inéluctable. Cette transition est rendue nécessaire par la nécessité de baisser drastiquement les émissions de CO2, mais aussi par l'importance, qui fait aujourd'hui consensus, d'un rééquilibrage de notre mix énergétique. Ce rééquilibrage doit permettre l'émergence de filières économiques fortes dans le domaine des énergies renouvelables, qui captent aujourd'hui la grande majorité des investissements énergétiques mondiaux. Dans le domaine électrique notamment,

les plus créatrices d'emplois et de développement local, mais pourrait aussi nous causer de grandes difficultés en cas de défaillance technologique des réacteurs actuels, lesquels, je le rappelle, sont tous peu ou prou du même modèle.

Nous voudrions insister ici sur quelques points qui nous tiennent particulièrement à coeur. Le groupe du RDSE est particulièrement attentif aux enjeux territoriaux, qui sont une des clefs de la réussite de la transition énergétique à mener- Nicolas Hulot l'a rappelé hier au congrès des maires. Nous voudrions ainsi tout d'abord, monsieur le secrétaire d'État, insister sur la question des territoires économiquement impactés par cette transition : ceux qui accueillent des tranches au charbon, dont le Président de la République a répété, à la tribune de la COP23, qu'il souhaitait les fermer avant 2021, ceux qui connaîtront la fermeture de sites nucléaires, ce qui ne concerne pas seulement Fessenheim, mais aussi- on y pense moins -les grands sites pétrochimiques, qui doivent dès aujourd'hui anticiper la fin des mobilités fossiles, du diesel et de l'essence. La Hollande vient d'annoncer la fin des véhicules thermiques pour 2030, la France l'annonce pour 2040 ; à ce développement désormais prévisible de la mobilité électrique s'ajoute la perspective d'une transition possible, le gaz, pour la mobilité des poids lourds. Tout cela conduit à une baisse régulière des activités de raffinage, c'est une évidence- il faut s'y préparer, il faut anticiper. Monsieur le secrétaire d'État, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler

si, comme en Loire-Atlantique, mon département, se trouve aussi au même endroit une centrale à charbon, des milliers d'emplois seront impactés, les coûts se comptant en centaines de millions d'euros pour les économies locales. Ces mutations sont inéluctables, mais doivent être anticipées de très loin. À ce titre, nous sommes très curieux de connaître la méthodologie que vous comptez développer pour sélectionner et, demain, accompagner financièrement ces territoires. Quant à tous les autres territoires, ils sont prêts, pour beaucoup d'entre eux, à s'engager dans cette transition, comme l'a montré le succès de l'appel à projet des TEPCV,

la parole de l'État dans le cadre des contrats déjà signés. Au-delà des TEPCV, la question de l'accompagnement de l'ensemble des territoires reste posée. Dans la loi relative à la transition énergétique et dans les lois de décentralisation,

Nous en avions d'ailleurs voté très majoritairement le principe au Sénat, l'année dernière ; il ne nous aura manqué que quatre voix à l'Assemblée nationale pour l'inscrire dans la loi. Mais nous comptons y revenir

j'insiste sur ce chiffre -, 12 milliards d'euros de recettes supplémentaires, ce qui n'est pas, là non plus, tout à fait rien. Nous vous alertons, monsieur le secrétaire d'État, sur un point : cette contribution ne sera pas payée

Or cette augmentation ne sera socialement acceptable que si nous avons les moyens, dans les territoires, d'augmenter l'offre de transport public ou d'accompagner les dispositifs nationaux de réhabilitation. Ainsi, l'affectation d'une part raisonnable de cette recette aux intercommunalités,

de la République a annoncé son désir de multiplier par deux les interconnexions électriques européennes, ce qui permettra de renforcer la sécurité globale du réseau. Cette évolution

Cette évolution annonce aussi probablement- mais cela, le Président de la République ne l'a pas dit -un accord historique entre la France et l'Allemagne, concernant les baisses parallèles du charbon et du nucléaire.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens d'abord à vous remercier pour l'occasion que ce débat nous offre d'aborder ce vaste sujet

de cette dernière. Je crois savoir que le Président de la République, le Premier ministre et le ministre d'État auront l'occasion, dans les jours ou semaines qui viennent, de préciser encore un certain nombre de points. Je sais combien la Haute Assemblée

C'est parler de ses relations internationales, européennes au premier chef- nous y reviendrons -, mais également mondiales, dans le cadre des négociations climatiques- vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur Dantec. Le discours du Président de la République, la semaine dernière, à Bonn, dans le cadre de la COP23, l'a encore illustré. Parler de l'énergie, c'est parler- vous l'avez dit -de nos territoires, de leur aménagement et de leur développement, de leur beauté, à travers la question des paysages, du littoral, du patrimoine. Et c'est parler des Français, qui règlent chaque mois leur facture de gaz et d'électricité, et paient, le cas échéant, le carburant pour leur véhicule ou le combustible pour leur chauffage. La politique conduite par le Gouvernement, et en premier lieu par le ministre d'État Nicolas Hulot, sous l'autorité du Premier ministre Édouard Philippe, se décline, sous tous ses aspects, selon deux principes simples : la prévisibilité et la sincérité. La prévisibilité est une condition absolue pour les acteurs du secteur, privés comme publics. C'est le sens de la programmation pluriannuelle de l'énergie, dont nous parlerons beaucoup en 2018- vous savez, mesdames, messieurs les sénateurs, que le Gouvernement souhaite associer le Sénat de manière très étroite à son élaboration.

Ce coût de la sincérité, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est le coût d'un investissement destiné à ce que nous construisions tous ensemble sur des bases solides. Le débat d'aujourd'hui- je vous remercie encore de l'avoir organisé -est ainsi l'occasion d'éclairer cette politique dans sa cohérence globale- c'est là le plus Commençons donc par le commencement, c'est-à-dire par la question des énergies fossiles. Le débat parlementaire sur le projet de loi Hydrocarbures se poursuit. Par-delà les divergences qui s'expriment, l'ambition de la France est claire : nous serons le premier pays au monde s'imposant à lui-même de laisser ses hydrocarbures sous le sol. du plan Climat, en juillet dernier, nous avions déjà annoncé notre intention de ne plus produire d'électricité à partir de charbon- j'aurai l'occasion d'y revenir. Cet engagement de la France a trouvé un écho sur la scène internationale avec la constitution d'une coalition pour la sortie du charbon, incluant le Canada et le Royaume-Uni. Enfin, cet engagement se décline concrètement dans l'accélération de la trajectoire carbone,

Ce sujet des énergies fossiles est indissociable de celui des transports, qui en sont les premiers consommateurs et représentent, excusez du peu, 40 % de nos émissions de gaz à effet de serre. Pour briser notre dépendance aux hydrocarbures, des solutions alternatives existent. Je pense naturellement au développement des véhicules électriques. Mais je pense aussi au gaz naturel pour véhicules, le GNV,

mais surtout d'imaginer des modèles de mobilité différents : intermodalité ou plateformes de partage en faveur des mobilités du quotidien, autant de solutions qui permettent de diminuer nos consommations de carburant. Vous l'avez compris,

De ce point de vue, les transports sont plutôt un exemple. Il ne suffit pas d'inventer de nouvelles sources d'énergie ; il faut aussi en consommer moins.

annoncera dans les prochains jours le début des concertations sur un plan majeur de rénovation thermique des bâtiments. Ce plan représentera un effort d'investissement de 9 milliards d'euros, intégré au grand plan d'investissement ; il s'agit d'une somme sanctuarisée, politiquement Le combat pour la maîtrise de notre consommation d'énergie se joue aussi dans l'innovation- je le disais à l'instant s'agissant des mobilités. Les champs ouverts par la révolution numérique sont immenses, qu'il s'agisse des transports- nous l'avons dit -, de l'autoconsommation, des réseaux intelligents, de l'effacement de pointe dans la gestion des réseaux électriques, avec pour ligne de mire la recherche sur le stockage. On le sait, le stockage de l'électricité est désormais le palier technologique, le noeud à franchir, qui déterminera le mix électrique

Pour le reste, la question posée est celle de la place de l'atome dans notre mix électrique. Cette question se pose à la France comme à tous les pays qui maîtrisent aujourd'hui l'énergie atomique. L'orientation de la loi de transition énergétique est maintenue nous ciblons toujours 50 % d'énergie nucléaire, mais à un horizon réaliste, sincère, disais-je, que nous définirons dans le cadre de la PPE, la programmation

le groupe de travail sur l'éolien, dont j'ai pris la responsabilité dans le cadre de la Conférence nationale des territoires, ou les Assises de l'économie de la mer, qui se déroulent aujourd'hui même, et au cours desquelles le ministre d'État évoque le sujet de l'éolien en mer- le Premier ministre s'est exprimé hier sur le sujet. Nous y travaillons et continuerons d'y travailler ; nous allons même accélérer. Monsieur le sénateur, vous y êtes revenu, ce débat sur l'énergie ne serait pas complet s'il n'abordait pas la dimension sociale du sujet. L'attention du Gouvernement, sur ce point, est constante et claire. Ainsi du plan Climat, qui prévoit la rénovation des « passoires thermiques » des ménages les plus modestes. Ainsi du paquet de solidarité climatique, qui comprend la généralisation du chèque énergie, la prime de conversion des vieux véhicules, élargie et renforcée pour les ménages non imposables, et ce de manière universelle, et l'évolution, prévue énergétique, en prime versée rapidement, qui facilitera l'investissement des ménages modestes. Cette attention constante se traduit également par la préoccupation du Gouvernement pour les territoires concernés par la transition écologique, et donc énergétique, et notamment par l'arrêt de la production d'électricité à partir de charbon, qui aura lieu pendant le quinquennat. À ce titre, nous engagerons, en 2018, la dynamique des contrats de transition écologique

Dans chacun de ces territoires, les contrats de transition comporteront un volet territorial et un volet destiné aux entreprises, ainsi qu'un volet social, dont l'objet sera précisément d'accompagner les salariés concernés par la transition écologique.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, quelles énergies pour demain ? Ce débat prospectif nous invite à réfléchir à la France que nous voulons léguer aux générations futures. Nos échanges sont d'une actualité brûlante : la COP23 a de nouveau dressé un constat alarmant sur l'urgence climatique, constat lui-même amplifié par l'appel récent de 15 000 scientifiques dans le journal. Nous ne pouvons plus attendre

Dès 1966, le général de Gaulle avait inauguré en Bretagne l'usine de la Rance, qui constituait une révolution à la fois technique et écologique. Depuis, rien sur ce sujet ! Début 2018, la société Tidal Lagoon Power inaugurera un projet prototype démonstrateur de lagon marémoteur d'une capacité de 320 mégawatts au large de la baie de Swansea, au Pays de Galles. Ce type de projet, s'il était développé le long des côtes françaises, en particulier de celles qui présentent un fort marnage, permettrait une production électrique équivalente, par lagon, à une demi-centrale nucléaire. En effet, des volumes d'eau très importants, deux fois par jour, tous les jours de l'année, conduisent à un résultat très régulier, très important pour être admis sur le réseau, fonction à la fois de la hauteur de la chute activant la turbine et de la superficie du lagon. Outre la production énergétique, la conception du lagon a vocation à protéger la côte et ses habitants contre les aléas climatiques ; elle améliore la gestion des crues et favorise les usages économiques locaux tels que la pêche ou l'aquaculture.

du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Elle estime toutefois que la France ne s'est pas dotée d'une visibilité à long terme pour ce qui concerne le financement de ces mesures.

décider, dans quelques jours ou quelques semaines, d'allouer à ces projets 75 millions d'euros supplémentaires, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2017. Restera néanmoins un déficit de 275 millions d'euros, qui manqueront à l'appel pour concrétiser les contrats qui ont été signés par ces collectivités. ces collectivités. Au moment même où le Président de la République déclare que le seuil de l'irréversible a été franchi et que les équilibres de la planète sont près de rompre, il est

demandera aux territoires concernés, c'est d'avoir commencé à engager le projet avant le 31 décembre 2017, ce qui n'est pas une nouveauté puisque cela figure dans la convention. L'État tiendra donc sa parole,

chers collègues, la France se fixe depuis plusieurs années maintenant des objectifs très ambitieux en matière de développement des énergies renouvelables. Ceux-ci ont été confirmés lors des différentes COP, mais aussi dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte en 2015, ainsi que dans le projet de loi mettant fin à la Le texte de 2015, voté par la précédente majorité, a introduit un nouvel outil de pilotage de la politique énergétique : les programmations pluriannuelles de l'énergie. Ces PPE Ces PPE concernent l'intégralité du territoire français : la métropole, mais aussi les zones dites non interconnectées, c'est-à-dire qui ne sont pas connectées au réseau électrique métropolitain du fait de leur éloignement ; je pense à la Corse et aux outre-mer. Les PPE sont le fondement d'une bonne gestion énergétique. Elles fixent et analysent les enjeux sur le sujet. Elles ont comme objectif global l'autonomie énergétique à l'horizon de 2030. Il y a quelques semaines, l'organisme qui gère le transport d'électricité, RTE, a publié son bilan prévisionnel accompagné de différents scénarios. Ce document va servir de base technique à la révision de la première période des PPE qui arrive à son terme l'année prochaine. Alors que la première période se concentrait sur le volet électrique, la prochaine période semble concerner toutes les consommations énergétiques. secrétaire d'État, quelles seront les priorités retenues et quel sera, dans les grandes lignes, le calendrier ? De plus, j'attire votre attention sur les zones non interconnectées. Du fait de leurs singularités géographiques, les PPE y sont coélaborées coélaborées avec les autorités locales pour s'assurer qu'elles sont adaptées à ces territoires. Parmi les caractéristiques de ces derniers, je cite pêle-mêle : les réserves d'énergies fossiles, les coûts de production plus élevés, plus d'ensoleillement, des sources d'énergie intermittentes. Ces atouts et ces faiblesses doivent être l'occasion d'innover en matière énergétique.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les enjeux de la transition énergétique sont des enjeux de société qui portent sur l'organisation des systèmes, sur nos façons de vivre, de produire et de consommer,

qui y aura accès ? Aujourd'hui, près de 8 millions de personnes sont en situation de précarité énergétique en France ; 2 milliards d'êtres humains sur les 7 milliards que compte notre planète- 10 milliards en 2050 ! -n'ont pas accès à l'électricité. L'énergie de demain doit être avant tout accessible à toutes et à tous. Nous croyons au développement des énergies renouvelables dans un mix énergétique. Cela demande tout d'abord de continuer à investir pour la sécurisation des centrales nucléaires, qui fournissement aujourd'hui près de 75 % de notre énergie, mais aussi dans la recherche et le développement pour le traitement des déchets. Il faut surtout investir massivement dans la recherche, le développement et la formation en matière d'énergies renouvelables de demain : géothermie, hydraulique, etc. Cela ne peut se faire, à notre sens, que dans le cadre d'un investissement public massif et de la création d'un pôle public de l'énergie, seul capable de réaliser les investissements dont nous récolterons les fruits dans vingt ans. Changer de modèle est coûteux et des investissements publics considérables sont indispensables. L'État, les collectivités locales doivent retrouver des marges de manoeuvre et de la capacité à se projeter dans le temps long. Or si le budget du ministère est en légère hausse, il s'inscrit toutefois dans une politique d'austérité, de baisse des dotations aux acteurs de cette transition et de renoncement à la lutte contre l'évasion fiscale, qui prive notre pays des moyens indispensables à cette révolution

Nous devons bâtir de toute urgence une vraie stratégie, réaliste techniquement, qui nous permette d'aller vers les énergies renouvelables. Cependant, les récents débats sur l'exploitation des hydrocarbures et les conclusions timides de la COP23 montrent combien les contraintes économiques sont souveraines. Les politiques que nous sommes, en tant que représentants des territoires, ont aussi le devoir de défendre les bassins d'emploi. Pour des milliers de salariés, transition énergétique est synonyme de reconversion professionnelle. L'emploi est l'une des variables clefs de la transition énergétique que l'on ne que l'on ne doit pas oublier. Nous ne pourrons avancer que si les stratégies de reconversion sont claires, accompagnées et anticipées par les pouvoirs publics. Ayant été moi-même élue dix ans à quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, je mesure combien un bassin entier peut être lié à une activité dominante.

le secrétaire d'État, est vertueuse, mais les régimes sont toujours un peu pénibles à mettre en oeuvre, nous le savons tous plus ou moins ... Qu'a-t-on prévu concrètement et rapidement pour accompagner tous les travailleurs concernés par ces mutations ? Vers quelles reconversions les orienter utilement,

Les énergies issues du vent, du soleil, notamment, ont une caractéristique, celle d'être variables et intermittentes, car elles dépendent des fluctuations de la météo. Autrement dit, ces énergies intermittentes produisent de l'électricité, mais pas forcément quand on en a besoin. Par ailleurs, elles peuvent saturer les réseaux lorsque des vents forts soufflent en même temps à l'échelle européenne. Or le fait de pouvoir stocker l'électricité permet de la restituer lorsque le besoin s'en manifeste, par exemple, lors des pointes de consommation. Le stockage permet donc de restituer l'énergie accumulée, en décalé, dans le temps, mais aussi là où se trouvent les besoins, c'est-à-dire dans un endroit différent du lieu où elle est produite. où en est-on du stockage de l'électricité ? On nous dit depuis longtemps que les solutions avancent. C'est très important, car cette nouvelle technologie conditionne un fort développement des énergies renouvelables qui sera rendu nécessaire, d'une part, par les comportements de plus en plus écoresponsables des consommateurs et, d'autre part, par la croissance massive de l'électromobilité dès lors qu'elle aura pris le pas sur l'essence et le diesel. Quelles sont donc dans ce contexte, les perspectives en matière de stockage ou de technologies nouvelles permettant de répondre aux enjeux actuels que sont, premièrement, une meilleure intégration des énergies renouvelables aux réseaux, lesquels devront répondre plus demain qu'aujourd'hui à une demande massive d'électricité avec le déploiement de l'électromobilité et, deuxièmement, une véritable sécurité d'approvisionnement électrique

du Rassemblement Démocratique et Social Européen. Ma question concerne le renouvellement des concessions hydroélectriques, ainsi que les perspectives du Gouvernement dans ce secteur. Lors de l'adoption de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notre pays s'est doté d'objectifs ambitieux en matière de développement des énergies renouvelables : celles-ci doivent représenter 40 % de la production d'électricité en 2030, alors que cette part s'élève actuellement à un peu plus de 20 %. L'hydroélectricité a un rôle important à jouer, la France étant le deuxième pays européen producteur avec environ 13 % de sa production totale d'électricité d'origine hydraulique. Cette source d'énergie, disponible à tout moment, s'inscrit pleinement dans la politique énergétique de notre pays ; il est primordial que l'État continue de garder la maîtrise sur cette production, qui participe à notre sécurité d'approvisionnement. Or la France fait aujourd'hui l'objet de démarches contentieuses concernant sa gestion du renouvellement des concessions hydroélectriques qu'elle a gelé depuis 2011, dont une mise en demeure par la Commission européenne en octobre 2015. Le régime des délais glissants, qui s'applique à de nombreuses concessions échues, est juridiquement très fragile. Il entrave la création de sociétés d'économie mixte instituées par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dont l'objet est d'exploiter des contrats de concession sur une vallée, afin de mieux associer les collectivités territoriales à la gestion des usages de l'eau, et de maintenir le contrôle public de l'État sur le parc hydroélectrique français comme sur l'ensemble de la production énergétique. Le retard pris dans le renouvellement des concessions hydroélectriques empêche également le perfectionnement structurel et fonctionnel du secteur, et engendre un manque à gagner considérable pour les collectivités territoriales et pour l'État lui-même, privés de la redevance prévue par l'article L. 523-2 du code de l'énergie. La Cour des comptes a évalué, dans un référé de 2013, que cette situation impliquera une perte de recettes cumulée de 600 millions d'euros d'ici à 2020 ; le département des Hautes-Pyrénées estimait pour sa part en 2015 à plus de 1,125 million d'euros le manque à gagner pour les collectivités territoriales concernées. Monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement prévoit-il d'engager rapidement le renouvellement des concessions arrivées à échéance, avec un éventuel dédommagement des collectivités lésées ? Enfin, quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour l'avenir et le développement de l'hydroélectricité dans notre pays ?

mes notes pour ne pas ajouter du trouble au trouble. La transition énergétique a notamment prévu la possibilité pour les collectivités locales d'être associées à la concession dans le cadre d'une société d'économie mixte hydroélectrique et a retenu l'option de regrouper des concessions hydrauliques hydrauliques liées, pour faciliter leur exploitation et favoriser la sûreté. Le statut des personnels sera préservé dans tous les cas et les cahiers des charges devront prévoir la reprise des personnels par le nouvel exploitant. Actuellement,

accord n'a pour l'instant été trouvé. Le Gouvernement compte poursuivre les discussions dans le même état d'esprit, à savoir en prenant en compte l'ensemble des enjeux et l'intérêt public. L'objectif est d'aboutir rapidement à une sortie du qui nuit aux investissements dans le secteur, suscite beaucoup d'inquiétude chez les élus locaux, et est source d'incertitude pour les entreprises et pour les salariés. La France continuera à défendre les regroupements de concessions, indispensables à la cohérence des vallées, les projets de prolongation, transmis à la Commission, ainsi que la possibilité pour EDF de participer au processus de mise en concurrence. La remise en concurrence est une politique nationale que nous souhaitons mener pour optimiser la gestion de nos barrages et relancer l'investissement, tout en redistribuant des ressources financières vers les territoires. Il ne faut pas oublier que les barrages appartiennent à l'État et que nous devons les valoriser ! La parole est à M. Pierre Cuypers, pour le groupe Les Républicains. Monsieur Monsieur le secrétaire d'État, la pollution de l'air tue prématurément 40 000 personnes chaque année dans notre pays. L'objectif de la France est d'instaurer un taux moyen d'émission de 95 grammes de CO2 par kilomètre parcouru pour les voitures neuves d'ici à 2020. Or, cette année, le Gouvernement baisse le seuil de 127 à 101 grammes pour les véhicules de société. Afin de le réduire davantage, le Sénat, dans sa séance du 16 novembre, a adopté un dispositif plus ambitieux au sein du projet Il a étendu l'exonération de la taxe sur les véhicules de société pendant une période de 12 trimestres aux véhicules fonctionnant au super-éthanol E 85, à l'instar du gaz naturel ou liquéfié, ce qui permet de répondre aux objectifs de réduction de CO2. La France a la chance d'avoir des carburants vertueux, qui réduisent notre dépendance énergétique. L'emploi du super-éthanol contribue à réduire les émissions de 65 % à 75 %. Alors, monsieur le secrétaire d'État, encourageons notre pays dans cette démarche.

Mais les Parisiens, contrairement à leurs voisins normands, ne pourront pas faire appel aux éoliennes. Le plan compte beaucoup d'actions, mais pas celle-là Le Gouvernement, de ce point de vue, a pris la mesure des enjeux, en faisant du développement des énergies renouvelables un axe de sa politique de transition écologique. Développer les énergies renouvelables, notamment l'éolien, c'est une ambition. Mais c'est aussi un impératif : veiller aux conditions de développement des entreprises à fort potentiel de ce secteur. Or, comme tous les secteurs, l'éolien a besoin de simplification, d'un cadre stable, qui s'impose à son activité. Je ne plaide évidemment pas pour l'abandon pur et simple des règles qui encadrent les énergies renouvelables en général, et l'éolien en particulier. Mais je partage la préoccupation du Gouvernement sur le bon niveau de contraintes pesant sur ce secteur. De manière générale, au-delà de l'éolien, favoriser les innovations technologiques en matière d'énergies renouvelables requiert un juste équilibre entre l'encadrement normatif et la souplesse pour encourager les initiatives.

quel est le périmètre exact de ce groupe de travail ? Où en sont les réflexions sur l'éolien terrestre ? Si propositions il y a, quelles seront les traductions législatives, réglementaires, budgétaires ou autre ? La parole

le secrétaire d'État, en France, l'hydroélectricité représente plus de 15 % de la production électrique nationale. C'est de loin la seconde source de production électrique derrière le nucléaire, la première source d'énergie renouvelable, ainsi que la seule source d'électricité renouvelable et stockable, en l'état actuel de la recherche. Dans le monde, en 2017, la puissance hydroélectrique est légèrement supérieure à 1 000 gigawatts, pour un potentiel estimé par l'Agence internationale de l'énergie à 3 700 gigawatts. C'est donc moins du tiers du potentiel hydraulique mondial qui est utilisé aujourd'hui. De fait, le développement de l'hydroélectricité dans le monde est en croissance constante pour des raisons objectives. C'est aujourd'hui le mode de production électrique le plus compétitif et le plus durable. Les barrages de type STEP- stations de transfert d'énergie par pompage -permettent à la Suisse de subvenir à nos besoins aberrants d'électricité de chauffage, lors des pics de consommation, les soirs de grand froid à Ces dispositifs, qui seront en 2030, selon l'ADEME, les seuls à permettre de stocker l'électricité de manière rentable, sont la fierté de l'entreprise GE Hydro de Grenoble.

La filière hydroélectrique possède une histoire riche à Grenoble et dans les Alpes. L'entreprise a toujours été en pointe dans ce domaine, et ce depuis de nombreuses décennies. Ce savoir-faire industriel centenaire a notamment contribué à la construction du barrage des Trois Gorges en Chine, le plus grand au monde. Pourtant, le Gouvernement n'a, pour l'instant, pas souhaité intervenir dans ce dossier, en refusant notamment d'entrer au capital d'Alstom, ou en rachetant les actions louées par Bouygues. Dans le même temps, le ministre de la transition écologique et solidaire annonce le report des objectifs d'évolution du mix énergétique pour la croissance verte, objectifs qui devaient être atteints en 2025, faute de solutions suffisantes en matière d'énergies renouvelables. Nous peinons à comprendre la stratégie industrielle du Gouvernement en matière de transition énergétique. Cette transition est pourtant urgente et indispensable pour respecter nos engagements de l'accord de Paris. en l'absence de grand débat national sur la transition énergétique qui semble pourtant indispensable, pouvez-vous éclairer la représentation nationale sur la stratégie du Gouvernement concernant le développement des énergies renouvelables en général et de l'hydraulique en particulier ?

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la stratégie nucléaire française est à la croisée des chemins ; c'est pourquoi elle manque de lisibilité. Voulons-nous sortir du nucléaire ou promouvoir un autre nucléaire ? Telle est la question fondamentale à laquelle nous devrons clairement répondre dans les années à venir. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte semble aller dans le sens d'une sortie du nucléaire, en fixant l'objectif de réduire sa part dans le mix électrique français à 50 % à l'horizon 2025. Mais même cet objectif intermédiaire va réclamer des efforts monstrueux. Je suis bien placé pour le savoir : un de mes proches est responsable du démantèlement de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux. Ce démantèlement dure depuis 25 ans et devrait prendre fin en 2100. Sur le site, 2 000 tonnes de graphite sont confinées dans des silos en attendant d'être enfouies, et 4 500 tonnes restent encore à extraire du réacteur. L'arrêt des centrales les plus anciennes va représenter un coût pharaonique. Dans ces conditions, envisager une sortie totale du nucléaire est sans doute utopique. C'est pourquoi la stratégie consistant à faire évoluer le nucléaire est plus que jamais d'actualité. C'est tout l'enjeu de l'EPR, mais c'est aussi l'enjeu de technologies révolutionnaires, comme la fusion, avec le projet ITER,

La parole est à M. Franck Montaugé, pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'énergie la plus propre est celle qu'on ne consomme pas, celle dont on n'a pas besoin. Et nous devons porter une attention particulière aux multiples façons d'économiser l'énergie. La transition énergétique s'appuiera pour beaucoup, on le constate déjà, sur les initiatives locales. À cet égard, plus de 500 territoires ont montré le chemin à suivre en s'inscrivant dès 2016, et à l'incitation très forte de l'État, dans le dispositif des territoires à énergie positive pour la croissance verte, ou TEPCV. Aujourd'hui, après s'être engagés auprès de leur population, de très nombreux maires, présidents d'intercommunalité et leurs conseils se voient contraints de renoncer à leurs projets d'économie d'énergie ou de production d'énergie renouvelable. Monsieur le secrétaire d'État, les maires et présidents d'intercommunalité qui se sont inscrits de manière exemplaire, fil des objectifs de la COP21 ne doivent pas être désavoués. Après une première circulaire envoyée aux préfets de région, très restrictive pour ce qui est de l'éligibilité des projets en cours, une seconde circulaire assouplirait les critères de sélection. Pouvez-vous nous l'exposer et rassurer les très nombreux élus qui montrent l'exemple de la responsabilité en matière de lutte concrète contre le réchauffement climatique ? La nécessaire évolution du mix énergétique de notre pays, du fait de la multiplication des points de production et d'injection de l'électricité sur les réseaux, transforme profondément notre modèle d'organisation, jusqu'ici centralisé, pour ne pas dire verticalisé. Ce phénomène nous oblige à penser, pour la partie liée à l'acheminement de l'énergie,

Notre-Dame-des-Landes est devenu le symbole des blocages auxquels sont confrontés beaucoup de nos grands projets. Qu'importe l'enjeu du projet ; qu'importe le processus décisionnel long et souvent minutieux qu'importent les procédures et les validations scientifiques ; qu'importe qu'un vote démocratique approuve le projet ! Partant du constat d'une France où les décisions publiques sont de plus en plus contestées,

présidée par Henri Cabanel, mission à laquelle j'ai eu l'honneur de participer, on peut tirer un certain nombre d'enseignements. Prenons l'exemple du développement de l'éolien en mer, qui, selon la loi, doit contribuer à hauteur de 40 % à la production d'électricité renouvelable à l'horizon 2030. Le premier appel d'offres a été lancé en 2011.

qui a été renouvelé après vingt ans de négociations et de procédures judiciaires, parce que les écologistes demandaient son démantèlement complet. Ma question est simple, monsieur le secrétaire comment l'État parviendra-t-il à faire appliquer des décisions publiques prises au terme de procédures d'expertises et de consultations publiques ? Comment, par entend-il concilier l'évolution envisagée du mix énergétique, pour plus d'énergies renouvelables, avec la difficulté liée à son acceptabilité dans la population ? Comment, enfin, conjuguer

Les collectivités territoriales auront désormais un rôle accru dans l'évolution de notre modèle énergétique. La gouvernance de l'énergie va évoluer en conjuguant les atouts d'un système très centralisé avec ceux des dynamiques territoriales telle est l'analyse du président de l'ADEME, que je partage entièrement. La loi NOTRe, en désignant les régions comme chef de file de la transition énergétique à l'échelon local, porte également, en filigrane, cette notion de territorialisation de l'énergie. Cependant, les acteurs locaux sont de plus en plus souvent à l'initiative de projets de production locale d'énergie, y compris participatifs, donc acceptés socialement. Mais ils se heurtent à des freins institutionnels ou administratifs de la part de l'État. Installer des turbines sur nos cours d'eau, des parcs photovoltaïques ou éoliens, ou valoriser la biomasse ne devrait plus s'apparenter un parcours semé d'embûches. Ces projets devraient être, au contraire, facilités. À un moment où les ressources des collectivités territoriales proviennent de moins en moins de l'État, il faut laisser

on comptera de quinze à vingt contrats démonstrateurs, il faudra prévoir l'adaptation des normes environnementales en la matière, puisque tous les acteurs locaux se seront mis d'accord, par voie de consensus en « mode Grenelle », sur les fiches-action et sur les projets qu'il convient de mettre en oeuvre sur le territoire. Dès lors, on peut très bien imaginer que l'autorité environnementale

à au moins 23 % la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique, contre 12 % en 2006. Parmi ces énergies renouvelables, la consommation de biomasse forestière, qui est la première ressource renouvelable en France, devrait ainsi passer de 9 millions de tonnes équivalent pétrole à plus de 13 millions dans la même période. Il est d'autant plus pertinent d'encourager les installations de cogénération utilisant la biomasse qu'elles sont riches en emplois locaux et par nature délocalisables. Elles participent ainsi au maillage territorial et à l'entretien des forêts. Par exemple, une centrale de cogénération installée dans mon département, voilà tout juste deux ans, a eu un fort impact local. Au-delà des mégawatts produits, elle a contribué à la création d'une centaine d'emplois directs et indirects en ayant recours à du bois récupéré, environ 100 000 tonnes par an, sur un rayon qui n'excède pas 50 à 100 kilomètres. Ce projet participe ainsi à l'entretien et à la régénération d'une forêt, qui gagne tous les jours dans nos montagnes des pans entiers de nos territoires, en raison de la déprise agricole. Pourtant, le rythme de développement de cette filière paraît insuffisant pour atteindre les objectifs. La compétitivité, comme vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'État, n'est toujours pas au rendez-vous. La concurrence du gaz naturel est forte et, face à celle des énergies fossiles, des volumes importants de bois ne trouvent actuellement pas de débouchés. Les tarifs d'achat sont insuffisants par rapport aux coûts de revient, en particulier pour les petites installations, qui sont pourtant celles dont l'impact en matière d'emploi et de bilan carbone est le meilleur. Le doublement du fonds chaleur n'est pas pour maintenant- j'ai d'ailleurs cosigné un amendement en ce sens avec ma collègue Nelly Tocqueville -et l'ADEME voit ses autorisations d'engagement diminuer dans le projet comment le Gouvernement envisage-t-il la place de la filière bois-énergie dans le programme de développement des énergies renouvelables, une filière qui a toute sa place, comme vous l'avez compris, monsieur le secrétaire d'État, dans nos territoires ruraux de montagne

du bois, il y a un enjeu de structuration de la filière. C'est absolument indispensable. La durabilité de la production d'énergie à partir du bois doit être évaluée. On ne va pas déforester pour ne produire que de l'électricité. Il faut être en cogénération et davantage utiliser les chutes de bois d'un certain nombre de métiers, de scieries, d'entreprises.

Le débat n'est pas simplement franco-français, vous le savez, il est naturellement mondial. Nous ne sommes jamais à l'abri d'un risque international, qui peut modifier singulièrement et fortement l'approvisionnement énergétique nous ne sommes pas à l'abri de l'apparition d'une nouvelle technologie ; nous ne sommes pas à l'abri de décisions politiques de pays étrangers, qui sont parfois nos partenaires. À cet égard, je veux évoquer le cas de l'Allemagne,

Ce développement, en particulier de l'éolien, aboutit à déstabiliser les prix de l'énergie électrique en Europe, puisque, vous le savez mieux que quiconque, monsieur le secrétaire

Mais on voit bien qu'on arrive au bout du bout de la logique sans accord de régulation, ou en tout cas d'entente, sur un coût du carbone commun à la France et à l'Allemagne. Cela fait partie des conversations que le Président de la République a avec Mme Merkel.

c'est vrai, à un moment donné, la PPE va devoir s'appuyer sur une visibilité du coût du carbone, parce que c'est celle-ci qui donnera la prévisibilité de notre trajectoire en matière d'énergie. Je crois que nous sommes convaincus de la même chose sur le sujet. À nous maintenant d'agir

qui ne connaît malheureusement pas le dynamisme de celle de l'éolien. L'énergie solaire est pourtant la plus compétitive, avec un prix qui peut descendre à 55 euros le mégawattheure, soit un coût nettement inférieur à celui de l'éolien. Si des parcs photovoltaïques sortent aujourd'hui de terre, je crois que nous devons aller beaucoup plus loin pour rattraper notre retard en la matière. Le projet de ferme solaire porté par la commune des Ponts-de-Cé, dans le Maine-et-Loire, est un bel exemple de ce qui peut se faire. Il s'agit de reconvertir une ancienne décharge en centrale solaire sur 13 hectares. Dommage qu'il ait fallu attendre huit ans avant que la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, ne valide le projet. Ne serait-il pas judicieux, monsieur le secrétaire d'État, de lancer une vaste opération de recensement des fonciers non agricoles qui pourraient faire l'objet de telles reconversions pour doper la filière ? Toujours en Maine-et-Loire- vous avez souligné tout à l'heure l'importance du côté participatif pour dynamiser certains projets -, les collectivités territoriales peuvent également compter sur une mobilisation citoyenne grâce à des associations ou des coopératives comme CoWatt ou Énercoop, qui se proposent d'accompagner les particuliers dans la transition énergétique. Cet engouement démontre que nos concitoyens sont prêts et attendent un soutien sans faille de l'État. Alors que les discussions concernant la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie portant sur la période 2023-2028 s'engagent, quelles sont, monsieur le secrétaire d'État, les mesures que vous envisagez pour encourager massivement la filière solaire en vue de rattraper nos voisins européens comme l'Angleterre ou l'Allemagne, pays pourtant nettement moins ensoleillés ? je vous remercie

qui ne proviennent pas d'un problème réglementaire, ce qui n'est pas le cas pour l'éolien, notamment l'éolien. Enfin, sur le foncier, j'ai prévu de sensibiliser les établissements publics fonciers pour recenser les friches, puisque, bien évidemment, sur des périodes données, dans le cadre d'un projet d'aménagement, dans les ZAC ou dans les concessions, utiliser ces friches pour produire de l'énergie est une solution qui peut être intelligente et intéressante, y compris pour celui qui possède le foncier.

en fixant dans une loi de programmation pluriannuelle de l'énergie le plafond par filière des nouvelles opportunités de production, ainsi que le plafond des surcoûts compensés aux opérateurs au titre de l'achat d'électricité issue de sources d'énergies renouvelables. Ma question est simple, monsieur le secrétaire d'État : le Gouvernement a-t-il aujourd'hui l'intention de proposer au Parlement de se prononcer sur ces sujets décisifs pour l'avenir économique du pays, notamment en lui permettant de prendre toute sa place et toute sa part ?

pour objectif le développement de la mobilisation et de l'utilisation de la biomasse, qu'elle soit forestière, agricole ou de déchets, en énergie, notamment pour atténuer le changement climatique, tout en respectant l'articulation des usages entre ses différents débouchés. Dès lors, la France possédant une importante ressource en biomasse, cette stratégie a également pour objectif de permettre une meilleure indépendance énergétique du pays et de tendre ainsi vers l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables en 2020 et de 32 % en 2030. malgré des initiatives convergentes offrant des perspectives au secteur de la biomasse, il semble qu'une véritable stratégie publique fasse défaut dans notre pays. En effet, la France ne dispose pas de réelle stratégie de bio-économie permettant de hiérarchiser les différents usages des ressources et de dépasser la question du partage de la ressource pour envisager les moyens de produire mieux et davantage. D'ailleurs, un rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de 2016 portant sur l'exploitation de la biomasse a rappelé les avantages associés à celle-ci à celle-ci : une énergie renouvelable dont la disponibilité est réputée permanente ; des ressources susceptibles d'être stockées ; un facteur de réduction d'émissions de gaz à effet de serre Ce rapport a souligné également le manque de vision globale à long terme et de stratégie publique pour une exploitation optimale de cette ressource. Enfin, l'exploitation de ces énergies est freinée par des lourdeurs administratives. Il faut en effet en France entre trois et quatre fois plus de temps que chez nos voisins italiens ou allemands pour obtenir les autorisations nécessaires. Depuis, un certain nombre de projets, je pense notamment à la transformation de la centrale à charbon de Gardanne, sont toujours en phase expérimentale. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous éclairer sur la façon dont vous entendez surmonter ces difficultés persistantes et faciliter la réalisation de projets de cette nature ?

la thématique des collectivités locales. Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le rôle des collectivités locales, l'avenir de la décentralisation et les suites à donner à la réforme territoriale ont un impact direct sur le quotidien des Français et sont autant de réponses aux fractures qui traversent notre société. Les enjeux futurs concernant ces thématiques sont donc très importants. De mon point de vue, ils se concentrent autour de quatre domaines : les relations entre l'État et les collectivités territoriales, les finances locales, les compétences des collectivités et l'achèvement de la modernisation de l'intercommunalité. En effet, les élus locaux sont légitimement préoccupés et inquiets du fait des incertitudes, qui pèsent très lourdement sur le devenir de leur collectivité. Or ils ont besoin de se projeter pour penser le futur de leur commune, de leur commune, car être élu aux côtés de leurs concitoyens, c'est, pour eux, se préoccuper de la gestion quotidienne, mais aussi être un bâtisseur d'avenir de leur collectivité. Cependant, comment agir si le flou l'emporte ?

? Avant de regarder plus précisément ces enjeux, il faut reconnaître que l'acte III de la décentralisation n'a pas eu lieu. Non pas parce que le précédent quinquennat n'avait pas la fibre décentralisatrice- le transfert aux régions de la gestion des fonds européens en est une illustration parmi d'autres -, mais parce que la priorité a été donnée à la modernisation de notre organisation territoriale. Je rappelle que notre pays compte, pour la première fois de son histoire, moins de 36 000 communes, grâce au succès du dispositif des communes nouvelles. Je rappelle aussi que la carte des régions métropolitaines a été redessinée, que la clause de compétence générale des régions et des départements a été supprimée et que le régime intercommunal a été rénové dans les grandes agglomérations avec la création des métropoles. Ce processus, alliant décentralisation de compétences précises et modernisation des structures, doit être poursuivi sans engager de nouveau big bang. Pour ce faire, il faut renouveler et institutionnaliser le dialogue entre l'État et les collectivités territoriales, c'est le premier enjeu. Un État décentralisé ne peut se passer d'une instance de discussion et de concertation pérenne réunissant l'État et les représentants des collectivités, où seraient discutés les projets de textes législatifs concernant ces dernières et mis sur pied un pacte de confiance.

À ce sujet, il faut noter que le projet du Président de la République d'exonérer 80 % des contribuables locaux de taxe d'habitation a eu un écho médiatique et populaire non négligeable pendant la campagne présidentielle. Cet impôt souffre effectivement de nombreuses lacunes et défauts et le projet a le mérite de cibler les classes moyennes et populaires. Il ne faut pas que cette exonération remette en cause l'autonomie fiscale des collectivités et finisse par se transformer en variable d'ajustement au sein des transferts financiers entre l'État, d'une part, et les collectivités territoriales, d'autre part. S'agissant des compétences, le Gouvernement doit être ouvert à de futurs transferts vers les collectivités, c'est le troisième enjeu. La suppression de la clause de compétence générale a permis de recentrer l'action des départements et des régions sur ce que j'appellerai leur coeur de métier : aux départements, les politiques de solidarité ; aux régions, les politiques structurelles, comme le développement économique ou la formation. Une décentralisation intégrale du service public de l'emploi vers les régions s'inscrirait ainsi en cohérence avec les compétences déjà exercées par les conseils régionaux. Le quatrième enjeu concerne l'intercommunalité. La refonte récente de la carte intercommunale et le renforcement progressif des compétences des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne doivent pas être perçus comme une remise en cause des communes,

qui est derrière l'affirmation des métropoles. Au moment où nous travaillons à une contractualisation de la relation entre l'État et certaines collectivités ou à la préparation de la deuxième réunion de la Conférence nationale des territoires, je veux ici témoigner de l'inquiétude, voire de la résignation- ce qui est souvent bien pire -, qui s'installe parmi les élus, les maires et leurs équipes. Les causes sont bien connues ; il s'agit en fait d'une succession de mesures rétrécissant toujours un peu plus le champ des libertés locales et affaiblissant le rôle des collectivités et des communes. C'est évidemment le cas avec les économies budgétaires de 13 milliards d'euros imposées au secteur local. Parce qu'elle intègre l'inflation et ne tient pas compte des efforts de gestion réalisés par les collectivités, cette mesure va rapidement se traduire par une baisse brutale des ressources et avoir des conséquences sur l'investissement. Même si, notamment lors du dernier quinquennat, un renforcement des mécanismes de péréquation a permis de réduire certaines inégalités entre collectivités ou territoires, la méthode de la contractualisation pour les plus grandes collectivités de notre pays est séduisante et beaucoup plus souple que la baisse de la dotation globale de fonctionnement, DGF, pratiquée sous les précédents mandats. Néanmoins, certaines des décisions préalablement annoncées ont été particulièrement mal ressenties, notamment dans les territoires ruraux et les banlieues

Ne faudrait-il pas, dès à présent, inscrire une clause de revoyure, afin de rassurer les élus et garantir le succès du dispositif de contractualisation ? En ce qui concerne les régions, si la carte territoriale a bien été remodelée, tout reste à construire. Tout autant que la taille ou le nombre d'habitants, ce sont les compétences, les capacités d'adaptation, y compris réglementaires, et la volonté de travailler en synergie qui comptent. La priorité de ces régions « XXL » sera désormais de redonner un sens à l'action qu'elles mènent sur l'ensemble de leur territoire, et cela grâce à une plus grande coopération territoriale. pragmatiques seront encouragées, je l'espère, chaque fois qu'elles permettront de renforcer la régionalisation. L'attribution d'une fraction du produit de la TVA en remplacement de la DGF va dans le bon sens, puisqu'elle renforcera l'autonomie fiscale des régions, tombée aujourd'hui à moins de 10 % ! Il faut faire confiance aux territoires et faire le pari de leur intelligence collective, de leur capacité à mener de grands projets. Il faut redonner du sens à la libre administration des territoires. C'est possible à Constitution constante. Les exemples de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna- cette collectivité a trois rois -, de la Corse, mais aussi de l'Île-de-France ou de Lyon le prouvent : la France est un État fédéral qui s'ignore

dans ce véritable big bang. La République s'est construite sur un triptyque hérité de 1789 : commune, département, Nation. La contre-révolution, parfois technocratique, bouleverse ce paysage

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis 2014, les conseillers métropolitains, tout comme l'ensemble des conseillers communautaires dans les communes de plus de 1 000 habitants, sont élus au suffrage universel par l'application d'un système de fléchage. Lors des débats entourant l'élaboration de la loi MAPTAM, le principe de l'élection de ces conseillers au suffrage universel dans le cadre d'un régime électoral autonome à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux a été retenu. Il a été convenu de renvoyer ce débat et les modalités de cette élection à une loi ultérieure. Celle-ci devait initialement intervenir avant le 1 janvier 2017.

la perspective d'une élection des conseillers métropolitains au suffrage universel direct dans le cadre d'un régime électoral autonome est perçue au sein des communes concernées avec une très forte inquiétude. Les maires ont démontré leur volonté d'accompagner les réformes votées par le Parlement, en s'associant pleinement à l'émergence des métropoles. Ils ont accepté d'exercer leurs compétences dans un cadre fortement élargi. Et ils ont aujourd'hui la légitime appréhension de se voir évincés par un système électoral, qui viendrait clairement dissocier représentation communale et métropolitaine. Dans un souci d'efficacité de l'action publique et de proximité avec la population, une telle entreprise ne semble pas souhaitable. Le groupe du RDSE avait d'ailleurs voulu, par voie d'amendement le 7 février dernier, acter l'abandon de cette hypothèse. de cette hypothèse. À la veille de l'ouverture du centième congrès des maires de France, M. le Premier ministre a rappelé par voie de presse que, dans ce débat, « tous les mécanismes qui remettraient en cause la place du maire ne [lui] semblent pas crédibles. » Madame la ministre, pouvez-vous nous éclairer sur la position de l'exécutif vis-à-vis de l'évolution du mode d'élection des conseillers métropolitains ? La parole

au congrès des maires de France. Vous avez rappelé vous-même que les conseillers métropolitains sont d'ores et déjà élus au suffrage universel direct, par fléchage

Les principes de libre administration et de non-tutelle d'une collectivité sur une autre ne permettent pas, en droit, de reprendre le modèle lyonnais pour les autres métropoles. Il importe par ailleurs que le mode électoral électoral retenu favorise la stabilité de l'assemblée élue et soit intelligible pour les électeurs. Aussi, à ce stade, le Gouvernement considère que le mode d'élection actuel, qui repose largement sur le suffrage universel direct, répond aux exigences juridiques et de démocratie citoyenne pour l'élection des conseillers métropolitains. Je pourrais d'ailleurs étendre mon propos aux autres intercommunalités,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite avoir des précisions concernant les emprunts toxiques, dossier qui inquiète encore localement. Je pense en particulier au cas de fusion entre plusieurs EPCI dans le cadre de la loi NOTRe et du schéma départemental de coopération intercommunale, lorsque l'un des EPCI avait précédemment souscrit un emprunt structuré. La loi a certes créé un fonds de soutien afin de permettre aux collectivités touchées par des emprunts structurés d'en sortir, condition de renoncer au contentieux engagé contre la banque. Certaines communautés de communes, bien qu'ayant reçu un avis favorable de l'État à l'octroi d'une aide du fonds de soutien, ont finalement préféré poursuivre le contentieux et ne pas donner suite à la proposition. Entre-temps, la fusion est intervenue puisque la loi NOTRe a imposé des regroupements d'EPCI au 1 janvier 2017, c'est-à-dire dans un délai très proche de la fermeture du fonds de soutien. L'emprunt structuré a ainsi été transféré dans le budget du nouvel EPCI.

Par ailleurs, ils ne peuvent plus faire appel au fonds de soutien, celui-ci ayant été fermé quelques semaines avant la création de ces nouvelles communautés, et alors qu'il restait encore 300 millions d'euros non consommés. Le Gouvernement a récemment annoncé : « la collectivité territoriale unique de Corse sera naturellement éligible au fonds de soutien destiné aux collectivités ayant souscrit à des emprunts toxiques [ ...] dans le cadre de la réouverture de ce fonds pour les collectivités issues de fusion. » Est-ce une disposition spécifique à la Corse ou d'autres collectivités ainsi que les EPCI sont-ils éligibles, comme le prévoyaient en 2014 les dispositions relatives au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risques ?

par l'article 31 de la loi de finances pour 2016. Pour bénéficier de ce fonds, les emprunteurs devaient déposer une demande d'aide avant le 30 avril 2015. Le Gouvernement examine actuellement les conditions de réouverture du fonds de soutien aux collectivités territoriales au regard des risques juridiques identifiés. En outre, cet examen approfondi nécessite une évaluation précise de la capacité de financement du fonds de soutien. En effet, une telle réouverture implique de définir précisément des critères objectifs, juridiques et financiers, justifiant la prise en compte des situations spécifiques concernant des collectivités ayant fusionné après

L'article 3 du projet de loi de finances pour 2018 instituant un mécanisme de dégrèvement de la taxe d'habitation est, d'abord, la traduction législative d'un engagement majeur du Président de la République, auquel le groupe La République En Marche souscrit. Voilà une mesure de justice sociale qui pose le premier jalon d'une refonte structurelle de la fiscalité locale sans amputer l'autonomie budgétaire des collectivités locales, par l'instauration corrélative de mécanismes de compensation. La taxe d'habitation, en l'état, est un impôt profondément injuste. Elle pose de réels problèmes d'équité fiscale entre les habitants des communes riches et ceux des communes plus pauvres, en particulier en raison des valeurs locatives qui demandent à être révisées depuis des décennies, qui ne l'ont jamais été. Globalement, elle frappe proportionnellement beaucoup plus durement les étudiants, les habitants des communes et quartiers populaires, ainsi que les personnes seules. En conséquence, sa suppression progressive peut être saluée, d'autant qu'elle s'accompagnera d'un gain de pouvoir d'achat significatif pour les Français : 10 milliards d'euros d'impôts en moins ! Cette réforme Cette réforme est pourtant devenue un élément de cristallisation du dialogue parlementaire : on en a extrapolé la portée financière vis-à-vis des collectivités, on en a déformé la logique d'action et on en a caricaturé la philosophie générale. Madame la ministre, peut-être ne serait-il pas inepte de rappeler aux membres de cet hémicycle et aux élus locaux qu'ils représentent que l'action de votre gouvernement a ceci de nécessaire qu'elle procède courageusement à la refonte d'un système qui, en l'état, galvaude l'autonomie fiscale ou financière

Mme la ministre. Monsieur Rambaud, vous avez rappelé l'engagement du Président de la République, l'aspect social de cette décision et, bien sûr, la garantie pour les collectivités territoriales de recevoir le montant

pallier la perte de recettes due au gel de la compensation ? Ensuite, qui payera au final ? Vous allez à juste titre me dire que ce sera l'État. Mais, dans l'État, quels sont les contribuables qui vont payer ?

baisse des dotations. La DGF reste stable. En ce qui concerne la taxe d'habitation, je souhaite revenir sur une question de vocabulaire : ce n'est pas une compensation, mais c'est un dégrèvement.

des impôts qui soient compris par nos concitoyens et justes pour les collectivités.

et nous pouvons relever des avancées notables sur différents aspects- régime indemnitaire, droit à la réintégration des maires et adjoints dans leur emploi à l'expiration de leur mandat, droit à la formation ...

Comme vous le savez, le Parlement, tout particulièrement le Sénat, a joué un rôle décisif dans la constitution progressive d'un réel statut de l'élu. Vous avez eu l'amabilité de rappeler que la dernière étape en date était la loi du 31 mars 2015, issue de

et le Président de la République lui-même a estimé que la fin du cumul des mandats était l'une des raisons fondamentales qui permettaient

vrai sujet. La parole est à M. Yannick Botrel, pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, débattre, même brièvement, de la question des collectivités peut être l'occasion d'une réflexion sur l'environnement dans lequel évoluent ces dernières. En ce sens, je veux centrer mon propos sur les relations entre l'État déconcentré et l'État décentralisé. Cette question des relations entre les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l'État est aussi ancienne que la décentralisation. de décentralisation mené à terme durant le quinquennat précédent, les élus locaux aspirent à une pause dans les réformes. Ces réformes ne sont pas encore pleinement appliquées, ne serait-ce que parce que le législateur a souhaité mettre en place des délais raisonnables d'application pour certaines dispositions. Il est nécessaire que les élus locaux disposent en ce sens, sur la durée de cette période, du soutien de l'administration déconcentrée. Or on note de la part du Gouvernement une volonté de recentrer le corps préfectoral selon une logique descendante. Plus qu'hier, le préfet se fait la voix du Gouvernement, ce qui fait partie de son rôle, mais ce qui ne saurait le résumer. Un renoncement au rôle de conseil des administrations déconcentrées pose un véritable problème, notamment en zone rurale. À cela s'ajoute également une problématique fondamentale : la décentralisation dans notre pays ne pourra se faire pleinement sans une réflexion, point par point, sur ce qui relève de l'État et ce qui dépend d'une ou plusieurs collectivités, dans chaque champ de compétences de la puissance publique. Il faut noter qu'il existe aujourd'hui, parallèlement au souhait de stabilité, une demande forte de meilleure coordination entre les politiques déconcentrées et décentralisées. Le Gouvernement semble s'engager dans une politique que l'on peut, à certains égards, qualifier de recentralisatrice. Je pense, pour ne prendre qu'un exemple, au pacte qui est proposé aux 319 plus grandes collectivités. Au-delà de l'intérêt apparent de cette solution, force est de constater que ce mode d'action, s'il paraît novateur, n'en est pas moins en rupture avec les pratiques passées de responsabilisation des collectivités et pourrait aboutir à une diminution de leur marge de manoeuvre en matière de conduite de l'action publique. La crainte existe donc que le Gouvernement ne fasse pas les choix qui devraient permettre de renforcer la décentralisation et l'efficacité des politiques publiques locales. Je vous remercie, madame la ministre, de nous éclairer sur ce point. La parole est à Mme la ministre. J'ai bien

des efforts déjà effectués, de l'évolution de la population, des caractéristiques socio-économiques et de la construction de nouveaux logements. C'est donc vraiment une politique qui se veut constructive entre l'État et les collectivités territoriales.

madame la ministre, mes chers collègues, les collectivités locales ne veulent pas de big bang territorial imposé d'en haut. Elles veulent au contraire être libres d'adapter leur organisation aux réalités locales, que ce soit par des fusions de communes, de départements, ou encore par l'approfondissement du fait métropolitain. les territoires, dans leur diversité, savent mieux que quiconque l'organisation qui est la plus pertinente pour eux. Depuis 2010, les collectivités territoriales ont été soumises sans cesse à d'importants changements du point de vue de leurs compétences ou de leurs structures, empêchant les élus de se projeter dans l'avenir avec sérénité, et ce d'autant plus que les collectivités ont également subi une baisse drastique des dotations versées par l'État, alors que lui-même était très loin d'avoir réalisé les économies qu'il leur avait imposées. Actuellement, les collectivités font face à deux évolutions avec la montée en puissance de grandes intercommunalités, de métropoles et le rôle nouveau dévolu aux régions. Cette période de mutation conduit à s'interroger sur le rôle et la place des départements et des communes, notamment en milieu rural. La commune, échelon de proximité, a montré qu'elle savait s'adapter aux changements de notre temps. C'est tout le sens de la « révolution silencieuse » des communes nouvelles, qui se sont orientées vers un vrai projet de territoire, voulu, partagé et non imposé par l'État Aujourd'hui, les collectivités veulent être mieux prises en compte, mieux associées à la prise de décision, mieux écoutées, mieux respectées. Madame la ministre, il faut faire confiance aux territoires, faire le pari de leur intelligence collective et de leur capacité à mener à bien les grands projets. Pouvez-vous nous assurer de votre volonté de retisser un lien de confiance avec les collectivités territoriales ?

ne veut pas faire de grande réforme territoriale pendant ce quinquennat. Il demande simplement à ses services sur le terrain, aux préfets d'accompagner

ont la capacité de mettre en place des politiques dont elles ont besoin, c'est-à-dire qu'elles ont la liberté de se saisir de compétences. C'est ce qu'on appelle la clause de compétence générale,

et Social Européen. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ma question concerne un outil bien connu des parlementaires et des élus locaux : la réserve parlementaire.

locale de 50 millions d'euros pour les collectivités et de 30 millions d'euros pour les associations. Je note à cet égard que, comparé au montant de la réserve pour 2017, le compte n'y est pas.

Tout d'abord, parce que je me souviens du décret du 20 juillet dernier ayant rendu les 260 millions d'euros de crédits DETR et DSIL pour l'exercice 2017. Ensuite, parce que la réserve parlementaire finançait en zone rurale de petits projets qui, souvent, n'étaient pas éligibles à la DETR. Enfin, parce que la composition et le fonctionnement de la commission départementale prévue à l'article L. 2334-37 du code ne sont pas satisfaisants. Il apparaît notamment que ces commissions sont, au mieux, des chambres d'enregistrement des décisions de la préfecture, et encore, seulement pour les plus grosses opérations. Nonobstant les améliorations que la navette parlementaire pourra apporter, le projet de loi de finances, je souhaite connaître les dispositions que vous entendez prendre pour améliorer

qui bénéficiaient souvent de la réserve parlementaire. La complémentarité entre la logique de déconcentration et la logique de décentralisation, qui caractérise la DETR, me semble tout à fait adaptée.

En outre, l'Assemblée nationale a abaissé à 100 000 euros le seuil de consultation de la commission. Évidemment, il faut aussi savoir que la DETR, comme la DSIL, la dotation de soutien à l'investissement local, qui a été pérennisée et qui sera inscrite dans le CGCT,

La mission qui m'a été confiée au sein de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation a consisté à suivre les différents textes de loi pour limiter à la fois le flux et le stock des normes.

adopté une résolution qui tendait à limiter le poids de la réglementation applicable aux collectivités territoriales. Nous avons également voté une proposition de loi constitutionnelle qui pose trois principes forts : pour une norme créée, deux normes supprimées le principe de prescripteur-payeur ; une interdiction de sur-transposition européenne. Et nous avons fait voter, à l'unanimité, une proposition de loi visant à simplifier les dispositions du code de l'urbanisme. Malgré les demandes répétées du président du Sénat, l'Assemblée nationale n'a jamais donné suite à cette requête, pourtant utile pour nos élus locaux. Madame la ministre, en cette période de diète financière pour les collectivités territoriales, à laquelle s'ajoute le coût normatif des textes de loi examinés en 2016, qui s'élève, selon le dernier rapport du CNEN, à 6,9 milliards

conclue le 23 juin 2016 entre le Conseil national d'évaluation des normes et le Sénat qui permet une coordination des initiatives prises en matière de simplification des normes. À titre d'exemple, le CNEN avait saisi le Sénat sur les difficultés rencontrées

Voilà donc un exemple de coopération particulièrement fructueuse. Plus généralement, la problématique de la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales s'inscrit dans le cadre du chantier de la Conférence nationale des territoires visant à une meilleure maîtrise du stock des normes. D'ores et déjà,

de cette règle au CNEN et montrer que le Gouvernement la fait strictement respecter. Le Gouvernement est décidé à aller plus loin. Le CNEN aura un rôle fondamental dans le processus, à la fois sur le flux et sur le stock. Il faudra, en particulier, lui donner une vision consolidée des projets de normes, afin qu'il puisse se prononcer en pleine connaissance de cause. Pour ce qui concerne l'urbanisme, le Gouvernement va présenter un projet de loi relatif au logement qui poursuit bien un objectif

l'État. Face à l'insoutenabilité de la dépense publique, face aux besoins d'efficience, le Gouvernement nous propose de relever ces défis collectivement. Il refuse la brutalité à l'égard des collectivités, il refuse la facilité, la baisse drastique des dotations- mieux, il les maintient ! Il fait le choix du courage, de la confiance et de l'intelligence collective. Le projet de loi de finances en est un signal. Le Gouvernement souhaite un pacte de confiance sur des orientations claires et qui ont été rappelées

générale, si quelques-uns sont sincères en manifestant leur inquiétude, d'autres la nourrissent avec une bonne foi relative. Cela pose la question du calendrier. Quand arriverons-nous au terme de ces réformes pour que chacun y voie clair et que les mauvaises langues s'arrêtent ?

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la teneur des questions posées aujourd'hui révèle l'immuable nécessité de faire part des doléances des collectivités locales. Il y en aurait tant à formuler ! Pour ma part, je concentrerai mon propos sur la complexité de la relation entre l'État et les collectivités locales. Comme vous le savez tous, contrairement à l'État, les collectivités sont soumises, dans la gestion de leur budget, à la règle de l'équilibre réel qui implique l'existence d'un équilibre entre entre leurs recettes et leurs dépenses, ainsi qu'entre les différentes parties du budget- sections de fonctionnement et d'investissement. Or, en parallèle à la gestion, différents transferts de compétences, toujours plus nombreux, sont réalisés.

a pire encore : elles sont pieds et poings liés et elles n'ont aucune visibilité sur l'avenir, aucune possibilité d'emprunter afin d'investir pour nombre d'entre elles, car elles n'ont aucune visibilité sur les dotations à venir de l'État, pas de calendrier fixe et pérenne. Elles n'ont également aucune vision sur les compensations : je pense, par exemple, à celles qui sont relatives à l'abattement de la taxe d'habitation, comme l'a souligné mon collègue Pascal Savoldelli. De plus, si les communes les plus denses disposent de moyens importants, notamment d'une administration étoffée qui leur permet de recueillir l'information plus facilement et ainsi d'anticiper, nombre de petites communes n'ont pas à leur disposition de cadres, ou simplement de personnels formés leur permettant de recueillir l'information sur les budgets à venir. Aussi, ma question est la suivante : quelles mesures concrètes et efficaces comptez-vous mettre en place pour améliorer la relation entre l'État et les collectivités et, dans un souci d'égalité de traitement, permettre à toutes les communes, quelle que soit leur taille, leur importance, d'accéder au même niveau d'information en provenance du Gouvernement, notamment en matière de dotation ou de compensation ? La parole est à Mme la ministre. Madame

Mme Corinne Féret, pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la Conférence nationale des territoires avait suscité des espoirs, qui ont aujourd'hui laissé place aux doutes. Les nombreuses mesures défavorables aux collectivités et aux territoires ont fini par affecter profondément la relation de confiance avec l'État. Les sujets de préoccupation s'accumulent, notamment depuis l'annulation de crédits dédiés aux quartiers et à la ruralité, la baisse des contrats aidés, ou encore l'atteinte majeure aux équilibres du logement social. De plus en plus, la perspective d'une contractualisation entre l'État et les plus grandes collectivités fait craindre un contrat unilatéral et non un engagement réciproque. On est bien loin de la démarche de décentralisation, conduite en France depuis François Mitterrand en 1981 Si les collectivités sont, bien entendu, favorables au rétablissement des comptes publics, elles s'inquiètent pour leur capacité à investir et à maintenir des services ou des équipements publics locaux de qualité. Sur le terrain, l'instabilité juridique et financière actuelle est source de préoccupation, tout comme la remise en cause du principe de libre administration des collectivités. Les élus déplorent également la stigmatisation dont ils font l'objet. Dire qu'il y a trop d'élus locaux en France et que ceux-ci ont un coût, comme l'a déclaré le Président de la République, c'est oublier que notre pays compte près de 580 000 élus locaux, dont une très grande majorité de bénévoles Personne ne peut nier dans cette enceinte le dévouement et la disponibilité de ces élus de terrain, de ces femmes et de ces hommes qui traitent des petits et des grands sujets de la vie locale dans nos villages, nos communes et nos quartiers.

que vous allez réduire le rôle des élus locaux, des maires au premier chef, en transférant à l'administration certaines compétences qui leur étaient jusqu'ici dévolues ? La parole est à Mme la ministre. Madame

madame la ministre, mes chers collègues, une fois n'est pas coutume, je veux remercier le ministre de l'intérieur du soutien qu'il a apporté aux élus qui sont allés manifester l'autre jour contre les prières de rue. Merci et surtout, madame la ministre, tenez bon

les territoires dans leur volonté de réforme et de développement économique. Nous espérons tous que la reprise économique permettra

que le ministre d'État, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb, a la même démarche que moi. Nous avons tous les deux été élu local et maire ; nous savons ce que sont les collectivités locales et nous ne pourrions pas, à notre poste, ne pas continuer la même politique de soutien aux collectivités locales.

les discussions budgétaires et les questions d'organisation, il se trouve que les collectivités locales constituent encore un sujet de débats et de passions. Pour ma part, je resterai très pragmatique en évoquant une problématique à laquelle sont confrontées les collectivités, qui restent bien souvent démunies face à cette mission. Il s'agit de la mise aux normes des bâtiments appartenant aux collectivités. Les élus souhaitent généralement répondre aux exigences et appliquer les principes émanant de différentes lois et aspirations : transition écologique,

peut-être pas très facile, mais il faut avancer dans cette voie parce que ce sera certainement moins contraignant. Par ailleurs, je rappelle que certains fonds,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'article 72-2 de la Constitution, à son alinéa 5, prévoit des dispositifs de péréquation le but est de gommer les écarts de richesses entre collectivités locales et, ainsi, de réduire les inégalités territoriales. En effet, comme vous le savez, tous les territoires ne sont pas également dotés ; ils connaissent des situations socio-économiques et géographiques fort différentes. À l'évidence, les territoires peu denses ne bénéficient pas des mêmes externalités que les métropoles, en termes d'infrastructures et de concentration de richesses. Si ces territoires ruraux sont capables d'innover, il arrive néanmoins qu'ils cumulent les handicaps, notamment géographiques.

Le législateur a progressivement mis en place des mécanismes de péréquation verticale et horizontale. Leur empilement a conduit à une certaine illisibilité ; ils gagneraient à être optimisés.

où l'on prive les territoires, notamment ruraux, de certaines ressources et où les collectivités les plus importantes sont appelées à poursuivre leur contribution au redressement des comptes de la Nation, comment imaginez-vous refondre le système de péréquation pour optimiser la solidarité territoriale, garantir un équilibre entre le monde rural, le monde périurbain et les métropoles et ainsi limiter les fractures territoriales ? Plus fondamentalement, sur quelle approche du développement territorial se fonderait cette refonte de la péréquation ? Choisirez-vous une métropolisation et un développement par ruissellement, si chers à votre gouvernement, ou bien préférerez-vous accompagner des dynamiques territoriales qui sont, elles, porteuses d'égalité ? La est à Mme la ministre. Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur le rôle joué par la péréquation dans la préservation des équilibres territoriaux, en particulier entre le monde urbain et le monde rural. me donne l'occasion de vous fournir quelques chiffres qui démontrent à quel point la péréquation, tant verticale qu'horizontale, bénéficie au monde rural.

perçoivent 34 % des ressources totales de ce fonds, alors que leurs prélèvements n'alimentent que 26 % de ces ressources. À l'inverse, les territoires urbains alimentent le FPIC plus qu'ils n'en bénéficient. C'est notamment le cas de la métropole du Grand Paris, qui fournit 34 % des ressources du fonds alors qu'elle ne bénéficie que de 4 % du reversement total. Au sein du monde rural, 10 000 communes bénéficient de la dotation de solidarité rurale cible. Il apparaît que 87 % d'entre elles sont bénéficiaires nettes au titre du FPIC et que 92 % d'entre elles ont bénéficié cette année d'une progression de leur DGF. Par ailleurs, je note que les petites collectivités rurales ne sont pas concernées par la démarche contractuelle de maîtrise des dépenses de fonctionnement qui est proposée dans le projet de loi de programmation des finances publiques. Avec les communes rurales, nous faisons donc le pari de la confiance

cette nouvelle attribution nécessite une ligne budgétaire, puisque l'entretien du patrimoine et les investissements- barrages, berges ou digues -incomberont dorénavant aux EPCI à fiscalité propre. Pour ce faire, nos élus locaux vont donc devoir trancher, comme d'habitude, entre deux options diminuer les dépenses, c'est-à-dire économiser sur certaines politiques publiques, ou augmenter les recettes, c'est-à-dire les impôts. À ce jour, la « taxe GEMAPI », même si elle n'est pas encore entrée en vigueur, est une composante de la taxe d'habitation et de la taxe foncière.

qui disposent de personnels formés et des compétences techniques nécessaires, est donc primordial. Néanmoins, un nombre important de communes ou de groupements s'appuient sur les associations syndicales autorisées, qui ont la connaissance du terrain, pour mettre en oeuvre la GEMAPI. Aussi voudrais-je savoir, madame la ministre, quel sort vous comptez réserver à cette catégorie d'associations. La parole est à Mme la ministre. Madame

qui est liée à la taxe d'habitation. Nous avons devant nous trois ans de tranquillité, si je puis dire, puisque la taxe d'habitation n'est pas supprimée, mais continue d'exister. Simplement, une partie des contribuables continue de la payer et, progressivement, l'État prend la place de certains autres. Nous n'aurons donc pas de difficultés pendant trois ans

Naturellement, la loi MAPTAM a préservé les compétences en la matière des syndicats et des associations syndicales autorisées ; il n'est pas envisagé de revenir

je fais le constat que la ruralité n'a toujours pas fait l'objet, à ce jour, d'un grand dessein national. Il y a aujourd'hui un impensé de la place des territoires ruraux dans l'avenir de la France. dans le contexte de mondialisation-globalisation que nous connaissons, notre pays a besoin de métropoles fortes et en développement ; c'est indispensable et vital ! Le rural que je suis en est convaincu et y contribue. Mais nous devons aussi penser la place des ruralités- la ruralité française est diverse et plurielle -en partant du principe, qui doit être un objectif politique partagé par le plus grand nombre, que les territoires ruraux et périphériques peuvent accueillir des populations et contribuer significativement à la création de valeur et de richesse nationale. Mme la ministre rappellera peut-être, à juste titre, les dispositifs qui existent au bénéfice des territoires ruraux, mais mon propos ne consiste pas à dire que rien n'est fait.

Ma question sera en réalité une proposition faite au Gouvernement : madame la ministre, l'État doit reconnaître les ruralités françaises et leurs habitants en engageant l'élaboration, largement participative, d'un projet de loi de reconnaissance et de développement des ruralités.

Monsieur le sénateur, comme vous le savez, je connais bien la ruralité, puisque j'y vis, et je suis sensible à vos propos.

proposée par le Gouvernement entre l'État, le préfet, et les collectivités locales. Cette contractualisation concerne exclusivement les 319 plus grandes collectivités de France, lesquelles sont à l'origine de 80 % de la dépense publique locale. L'État leur demande,

Madame la ministre, vous avez déclaré que cette contractualisation serait un « travail de dentelle » qui prendrait en compte différents critères, comme la taille de l'agglomération, l'évolution de sa démographie ou l'importance des charges de fonctionnement. si cette contractualisation est aussi technique à établir, pourquoi ne pas l'avoir proposée de prime abord à l'ensemble des collectivités locales pour déterminer un barème national, plutôt que d'en réserver le périmètre aux seules communautés d'agglomération de plus de 150 000 habitants, ainsi qu'aux communes de plus de 50 000 habitants Cette contractualisation exclut les villes moyennes, les petites communes et les villages. Elle envoie un très mauvais signal à ces territoires tout en renforçant l'inquiétude budgétaire et le sentiment d'abandon des élus qui les représentent. De plus, dans le cadre de ce contrat proposé aux grandes collectivités locales, certaines d'entre elles n'ont pas toujours été vertueuses ces dernières années. Comment ne pas voir dans la contractualisation, pour les collectivités les plus dispendieuses, un effet d'aubaine, puisqu'elles se raviseront dans leur gestion ? Les collectivités locales qui ont choisi d'être vertueuses depuis longtemps, car elles sont gérées par des élus responsables et courageux, seront également désavantagées, puisque leurs efforts passés ne seront pas récompensés. Pourtant, ces collectivités ne méritent pas cette menace d'assèchement fiscal. Madame la ministre, comptez-vous mettre en place un dispositif mesurant les efforts et les économies déjà consentis dans le passé, et non pas seulement à la date d'effet du contrat, afin de ne pas soumettre ces collectivités à une double peine budgétaire ? est à Mme la ministre. Madame la sénatrice, le contrat de mandature entre l'État et les collectivités locales repose effectivement sur la confiance. de loi de programmation des finances publiques définit un cadre et des objectifs, mais la méthode pour y parvenir sera laissée à l'appréciation de chaque collectivité. Telle est la philosophie du pacte de confiance que nous entendons nouer entre l'État et les collectivités.

En 2010, le Gouvernement décidait la suppression de la taxe professionnelle au motif que les éléments servant à son calcul étaient anti-économiques. Il en est résulté une perte de 13 milliards d'euros, qui a été compensée dans les conditions que vous savez. vous nous proposez la suppression de la taxe d'habitation. Non ! Cela permettra peut-être d'améliorer le pouvoir d'achat des familles, mais on aurait pu faire un autre choix que celui d'obérer les marges de manoeuvre des communes.

de la Constitution, sera en tout état de cause respectée. La réforme de la taxe d'habitation n'altère pas le ratio d'autonomie ainsi défini. En effet, la taxe d'habitation n'est pas supprimée simplement l'objet d'un dégrèvement, et non pas d'une exonération. La dynamique des bases reste donc acquise à la collectivité et la taxe d'habitation dégrevée demeure une ressource propre au sens de la Constitution.

Comme vous, je suis convaincu que l'intercommunalité représente une chance de survie pour les communes et je reste pleinement conscient que la mutualisation des moyens humains et financiers est un enjeu déterminant, notamment en milieu rural. En revanche, il est certain que l'intercommunalité doit impérativement être consensuelle et cohérente pour servir d'outil en faveur d'un projet de territoire. Quelle est la logique actuelle ? Une course aux collectivités « XXL », coûteuses et peu démocratiques

Fruit d'une vision dogmatique de la loi NOTRe qui consiste à concentrer les compétences sans s'interroger sur l'opportunité ou la faisabilité d'un tel transfert, la disposition actuelle dépossède les élus ruraux de tout choix, qu'ils ont souvent déployé des solutions adaptées à la géographie et à la morphologie des territoires. L'enjeu est d'améliorer la gestion de ces politiques en redonnant pouvoir de décision et de responsabilité aux élus locaux. L'idéologie consistant à « éplucher » les compétences des communes pour les affecter sans choix aux intercommunalités se heurte à une réalité concrète : le périmètre des nouveaux EPCI ne correspond pas nécessairement aux périmètres des syndicats gérant ces enjeux. L'enjeu est aussi économique, puisque, dans de nombreux cas, le coût du transfert à l'échelon de l'intercommunalité se répercutera sur le prix de l'eau. En d'autres termes, le maintien du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement à l'intercommunalité serait la preuve de la poursuite d'une vision technocratique. La parole